La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 18 mars 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation Le procès-verbal est adopté. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Par ailleurs, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi

à étudier la possibilité d'une mise en cohérence de sa politique énergétique avec ses ambitions écologiques, présentée par M. Bruno Retailleau, Mme Sophie Primas, M. Daniel Gremillet et plusieurs de leurs

débattre au Sénat de cette proposition de résolution invitant le Gouvernement à étudier la possibilité de mettre en cohérence sa politique énergétique avec ses ambitions écologiques.

De toutes les sources d'énergie, c'est la moins émissive : en effet, les émissions d'une centrale nucléaire sont limitées à 6 kilogrammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. C'est une filière d'excellence,

Qu'on se le dise, l'énergie nucléaire est garante de l'égalité dans l'accès à l'énergie, sur tout le territoire de la République ; elle est aussi garante de la place de l'État dans le secteur de l'énergie face aux pressions concurrentielles et d'un faible coût de l'énergie, primordial pour le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de nos entreprises. La production d'énergie nucléaire est, en France, un service public, une mission régalienne, qui conditionne tout à la fois notre vie sociale, notre activité économique et notre transition écologique. Notre souveraineté et notre efficacité énergétiques en dépendent. Face à l'urgence climatique, c'est grâce à cette source d'énergie que nous pouvons réduire durablement nos émissions : la décarbonation de notre économie passe par l'énergie nucléaire. Parce que je crois en l'avenir de la filière nucléaire, je suis préoccupé par la politique énergétique conduite par le Gouvernement. Si le Sénat a adopté la loi Énergie-climat en 2019, c'est parce qu'elle comprenait plusieurs avancées significatives pour cette filière : le report de dix ans de la réduction à 50 % de la proportion d'énergie nucléaire ; la prise en compte de l'inflation dans les ressources perçues par EDF cadre législatif pour l'hydrogène bas-carbone, produit à partir de l'énergie nucléaire. Or le Gouvernement n'a cessé de décevoir depuis lors. En effet, nous avons assisté à l'arrêt du démonstrateur de réacteur à neutrons rapides Astrid, en 2019, et des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, en 2020 : c'est regrettable, d'autant qu'aucune raison de sécurité Par ailleurs, sur les 110 milliards d'euros du plan de relance, seuls 200 millions d'euros sont alloués à l'énergie nucléaire, alors qu'elle représente les trois quarts de notre mix énergétique. Les réformes en cours du marché de l'électricité, à commencer par celle régulé à l'énergie nucléaire historique (Arenh) et le projet de réorganisation « Hercule » au sein d'EDF, sont conduites dans une opacité inacceptable. C'est pourquoi je me félicite de ce que la commission des affaires économiques du Sénat, à défaut d'être associée à ces réformes, comme elle l'avait demandé, ait de son propre chef institué un groupe de suivi pluraliste. En outre, le ministère de la transition écologique a commandé à Réseau de transport d'électricité (RTE) et à l'Agence internationale de l'énergie (AIE) un scénario « 100 % renouvelables » d'ici à 2050. C'est une entorse faite à la loi quinquennale, prévue par la loi Énergie-climat, qui détermine seule, en principe, l'évolution de notre mix énergétique après 2023. Je veux dire très clairement ici que le non-respect par le Gouvernement de la loi quinquennale est inadmissible. Totalement ! Outre Outre ce scénario, je rappelle que le Gouvernement a voulu supprimer l'évaluation de la loi quinquennale, à l'occasion de la loi de finances pour 2020. Aujourd'hui, il souhaite revenir au décret pour la détermination d'objectifs en matière de certificats d'économie d'énergie, mais aussi en matière d'énergies d'énergies renouvelables, dans le cadre notamment du projet de loi Climat et résilience. La pandémie de la covid-19 a des répercussions très importantes sur la filière nucléaire. Dans son bilan électrique pour l'année 2020, RTE a relevé que, « du fait de la pandémie de covid-19, l'année 2020 marque une rupture ». Au total, on observe une chute de 3,5 % de la consommation d'électricité, 7 % pour sa production et 18 % pour son prix : c'est considérable ! Cette crise affecte au premier chef notre fournisseur historique, EDF, avec une chute de la production d'énergie nucléaire de 13 %, une perte de recettes de 2 milliards d'euros et un décalage du programme d'« arrêts de tranches », c'est-à-dire les opérations de maintenance des centrales nucléaires. Cette crise pèse sur notre sécurité d'approvisionnement. Sur ce point, RTE a relevé que notre production d'électricité sera « sans aucune capacité supplémentaire » jusqu'en 2023. Cette crise éprouve notre souveraineté énergétique. Selon RTE, la France a été importatrice d'électricité pendant quarante-trois jours en 2020, contre vingt-cinq en 2019. Enfin, cette crise érode notre capacité d'investissement. EDF est ainsi confrontée à un « mur d'investissements ». Grevé d'une dette de 40 milliards d'euros, le groupe doit parvenir à financer le « grand carénage », les chantiers des EPR, mais aussi ses programmes d'énergies renouvelables. Dans ce contexte très perturbé, les réponses apportées par le Gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux de la filière nucléaire. Tout d'abord, la chute de la production d'énergie nucléaire résulte non seulement d'un facteur exogène, la crise de la covid, mais aussi d'un choix politique, la fermeture de la centrale de Fessenheim. C'est un immense gâchis ! Sur le plan économique, tout d'abord, cette fermeture coûte 5 milliards d'euros. Sur le plan social, ensuite, 150 salariés ont déjà quitté le site et seuls 60 resteront à terme. Sur le plan énergétique, enfin, le parc nucléaire a perdu 1,8 gigawatt de puissance. Face aux difficultés liées à la sécurité d'approvisionnement, la ministre Barbara Pompili et la secrétaire d'État Bérangère Abba se sont contentées d'appeler, ici même, « à diversifier notre mix énergétique C'est une erreur majeure, car les énergies renouvelables, intermittentes, ne permettent pas de surmonter « la pointe de consommation » hivernale. En clair, si nous délaissons nos centrales nucléaires nationales, nous ferons tourner à plein régime les centrales à charbon étrangères. Loin de veiller à notre souveraineté énergétique, le Gouvernement n'offre pas de solutions pour le retour des turbines nucléaires, fabriquées par Arabelle, ou l'avenir des services nucléaires, assurés par Endel.

le Gouvernement ne propose aucune réponse à ce jour. La réforme de l'Arenh est conditionnée au projet « Hercule », la construction de nouveaux EPR à la mise en service de celui de Flamanville, les investissements mobilisables aux négociations sur la « taxonomie verte ». Dans le domaine du nucléaire, tout est en chantier, tout est en suspens. Aucune décision n'est prise, aucune information n'est donnée. Les réformes sont tantôt imminentes, tantôt encalminées. Or il devient urgent que le Gouvernement s'exprime, qu'il affirme un cap nucléaire, clairement établi et vraiment appliqué. À quelques semaines de l'examen par le Sénat du projet de loi Climat et résilience, cela devient une nécessité. Aucune disposition de ce texte n'évoque le nucléaire. C'est tout à fait paradoxal, mais peut-être aussi très révélateur Au-delà de ce constat, très inquiétant, que faire ? J'ai la conviction que le moment est venu de réaffirmer notre confiance en la filière nucléaire : un cap, des projets, des financements. Nous devons, tout d'abord, fixer un cap ambitieux. Dès l'examen de la loi Énergie-climat, j'avais alerté sur l'insuffisante évaluation préalable de la fermeture des quatorze réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Nous en mesurons aujourd'hui les conséquences pour les territoires et les salariés concernés, dans le contexte de crise de la covid-19.

Face à un exécutif hésitant, le Parlement doit jouer tout son rôle : je plaide pour que la prochaine « loi quinquennale » soit celle d'une politique nucléaire ambitieuse. Nous devons, de plus, promouvoir des projets. Cela suppose de redoubler d'efforts pour sortir des difficultés du chantier de l'EPR de Flamanville, a imputées à une « perte de compétences généralisée ». Les difficultés de la filière nucléaire sont à l'image de celles de l'industrie : notre pays s'est trop longtemps résigné à une perte d'emplois, de compétences ou de technologies, sous l'effet de la mondialisation des échanges. Cette période est révolue, et il nous faut renouer avec le volontarisme : la réindustrialisation de la France commence par la renaissance de la filière nucléaire. À cette fin, un effort de recherche et d'innovation suffisant doit être consenti, en direction notamment des petits réacteurs modulaires, des réacteurs à neutrons rapides et des électrolyseurs à hydrogène bas-carbone. Par ailleurs, des choix clairs doivent être faits : le projet de construction de trois nouvelles paires d'EPR, proposé par EDF, mérite d'être étudié avec attention. Enfin, nous devons mobiliser des financements suffisants. Cela implique de rehausser les ressources nécessaires dans le cadre du plan de relance, de défendre l'énergie nucléaire dans les négociations sur la « taxonomie verte » et de préparer l'évolution de l'Arenh après 2025. Au total, nous attendons du Gouvernement un changement de politique, pour redonner à l'énergie nucléaire la place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. La France a besoin d'une colonne vertébrale énergétique. Je souhaite que l'examen de cette proposition de résolution soit l'occasion de rappeler l'attachement du Sénat à l'énergie nucléaire,

reconquérir la production industrielle de notre pays et garantir l'accessibilité à tous nos concitoyens. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter la proposition de résolution qui vous est soumise aujourd'hui. La parole

La politique publique énergétique de notre pays est affectée par l'indécision du Gouvernement. Toutefois, il ne s'agit pas uniquement de son incapacité à définir un scénario réaliste. Le Gouvernement dispose en effet de tous les moyens et données pour établir des scénarios plausibles s'agissant de l'évolution de la consommation énergétique, notamment électrique. Ainsi, nous le savons, entre 2012 et 2019, la consommation énergétique finale n'a diminué que de 1,4 %, alors que le plan pluriannuel de l'énergie 2016 prévoyait une baisse de 12,3 % entre 2012 et 2023.

Cela ne paraît pas très sérieux. La réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 est une hypothèse irréaliste. C'est un mirage sur lequel ne peut pas reposer une politique énergétique honnête et juste.

Mais gouverner, c'est autre chose, c'est faire des choix. Il ne s'agit pas de promettre et de faire croire ; il s'agit de faire ! L'une des premières responsabilités du Gouvernement est ainsi d'éviter les risques de carences, de coupures d'approvisionnement électrique ou, pire, de blackout énergétique- nous en avons débattu ici la réalisation de ces scénarios catastrophes à court et moyen termes, il n'y a pas d'autres choix que de se fonder sur les moyens dont dispose la France, ce qui suppose d'accorder une place centrale au nucléaire, qu'on le veuille ou non, dans notre bouquet énergétique. Pour réaliser ses ambitions écologiques, la politique énergétique du Gouvernement doit aussi gagner en clarté. En ce sens, la mise en concurrence des concessions hydrauliques, sous la pression de la réglementation européenne, et le projet Hercule ne sont pas des bases solides. D'une part, elles portent atteinte à la souveraineté énergétique nationale ; d'autre part, elles négligent la diversification de notre mix énergétique. L'hydroélectricité peut évidemment concourir à atteindre l'objectif de « neutralité carbone » en 2050, mais pas à n'importe quelles conditions. J'interrogeais récemment encore, ici même, la ministre de la transition écologique à propos de la prorogation des concessions des barrages du Lot et de la Truyère en Aveyron, qui représentent 10 % de l'énergie hydroélectrique en France ; aucune réponse claire ne m'a été donnée. Le problème est donc celui d'une invocation idéologique de la transition écologique, qui se décline dans tous les domaines des politiques publiques, de manière bien souvent irresponsable. Récemment encore, le Gouvernement a pris des mesures contradictoires avec ses annonces passées concernant la filière automobile diesel, en décidant ne plus soutenir la transition écologique de cette filière. les conséquences se répercutent en cascade, avec des licenciements en nombre : plus de 1 000 suppressions d'emplois en Aveyron, dans les usines Bosch de Rodez et SAM de Viviez, et des territoires désabusés. Je pourrais également évoquer l'impact économique de la réglementation environnementale RE 2020. Sur ce sujet, les mêmes causes produisent encore les mêmes conséquences manque d'association des professionnels, insuffisance de l'évaluation réalisée et, surtout, crainte des ménages face à l'augmentation des coûts induits par ces mesures. Le renforcement de l'efficacité énergétique des logements neufs est nécessaire, mais sa mise en oeuvre est à revoir. En évoquant ces problèmes, je ne m'écarte pas du sujet de la présente résolution. Au contraire, je montre à quel point cette résolution est pertinente est pertinente : en effet, sur bien des sujets, la transition écologique est invoquée par le Gouvernement pour justifier des choix incohérents, irréalistes et au final néfastes pour nos concitoyens, pour leur portefeuille et pour l'aménagement du territoire. Les citoyens ne sont pas dupes. Ils nous font part de leurs inquiétudes et de leurs préoccupations, comme aujourd'hui, en Aveyron, à Onet-le-Château ou à Viviez. Ils dénoncent l'incohérence des choix gouvernementaux sous couvert d'ambitions écologiques. La mise en cohérence de la politique énergétique, conciliée avec des ambitions écologiques fortes, est une nécessité sur laquelle la responsabilité du Gouvernement doit être affirmée. Il est urgent de poser les jalons d'une véritable politique énergétique pluridimensionnelle dans laquelle le nucléaire a toute sa place.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la neutralité carbone à l'horizon 2050 : oui, mais comment ? Il est juste de s'interroger sur les moyens pour l'atteindre, comme le fait cette proposition de résolution. Le principal objectif est ainsi de sortir des énergies fossiles polluantes et de développer les énergies non émettrices de gaz à effet de serre. La stratégie française doit composer avec des impératifs climatiques et viser l'indépendance énergétique. La composition de notre bouquet énergétique en constitue un aspect. Il faut ainsi travailler à des évolutions pertinentes pour le rendre à la fois sûr, décarboné et compétitif. Je pense que l'une des clés de la réussite est d'augmenter la part de l'électricité dans notre mix énergétique. La décarbonation de secteurs entiers de notre économie sera un élément crucial, et la priorité doit donc selon moi aller vers les secteurs industriels fortement émetteurs, comme l'acier, le ciment et les transports. Les demandes augmentent et les émissions doivent baisser. Si nous parvenons à décarboner ces secteurs, l'effet d'entraînement sera immense. L'énergie nucléaire, fleuron de l'industrie française depuis les années a le mérite d'apporter une solution à la décarbonation de notre mix énergétique, comme l'a fait remarquer Brice Lalonde. C'est un atout à préserver, comme le souligne la proposition. C'est le point névralgique du débat électrique en France. Cependant, plusieurs problèmes se posent. Premièrement, il faut préserver et développer notre savoir-faire reconnu en la matière et poursuivre les innovations technologiques, qui nécessiteront de lourds investissements. C'est une question d'économie et d'emplois. Le secteur place de grands espoirs dans le nucléaire de quatrième génération, qui pourra fonctionner avec certains déchets.

et sécurité nationale. En effet, toutes ces installations peuvent représenter des cibles privilégiées pour les terroristes. Si le nucléaire est le coeur du débat électrique, alors les énergies renouvelables en sont les poumons. Si le nucléaire est indispensable dans notre mix énergétique, les énergies renouvelables sont tout aussi cruciales. La diversité des sources d'énergie est stratégique ; elle apparaît comme un choix de bon sens. Les énergies renouvelables deviennent de plus en plus efficaces. Elles sont aussi de moins en moins onéreuses et concurrencent aujourd'hui les prix du nucléaire. L'électricité en France représente déjà une part importante du budget pour de nombreux ménages ; la précarité énergétique doit continuer de reculer. Le solaire doit également retenir toute notre attention. Les progrès déjà réalisés dans ce domaine sont immenses et la technologie avance à pas de géant- je pense notamment au taux de recyclabilité des panneaux solaires. Par souci de compétitivité, les futurs investissements dans ce secteur, comme dans celui des batteries ou de l'hydrogène, doivent être réalisés à l'échelon européen, d'autant que, dans ce domaine, nous dépendons fortement des fournisseurs asiatiques. Bien sûr, j'ai lu dans la proposition de résolution toutes les craintes autour de l'intermittence des énergies renouvelables et de leur stockage. Là encore, je crois que les innovations technologiques sont d'ampleur et que les solutions sont désormais à portée de main. Nous devons poursuivre inlassablement le travail et les investissements afin de permettre l'émergence de solutions nouvelles, comme celle qu'apporte l'hydrogène, la conversion d'électricité en gaz. La part d'électricité dans notre bouquet énergétique et la baisse des émissions sont directement liées aux usages des consommateurs. Il faut poursuivre notre action, notamment dans les performances thermiques de l'habitat et dans le secteur automobile.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, abandonner les énergies fossiles est une urgence, un impératif de survie pour l'humanité Produire notre électricité de demain sans émettre de CO2 est indispensable, même si, rappelons-le, 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de secteurs sans aucun lien avec la production d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant. Les choix politiques effectués sur les questions énergétiques engageront la France pour des décennies, voire, selon les décisions, pour des millénaires. Pour y répondre, deux options sont sur la table. La vôtre une relance du nucléaire, cette énergie obsolète, ... Non ! ... fragile, dangereuse, chère, qui oblige l'État à une nationalisation du parc nucléaire pour assurer la charge des investissements colossaux. La nôtre : un engagement immédiat, massif et sans faille dans la sobriété énergétique et les énergies renouvelables, avec parallèlement une sortie programmée du nucléaire. À l'heure où les choix du Gouvernement s'orientent vers la décision irresponsable de construire un nouveau parc nucléaire EPR en France, il est temps d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une énergie d'avenir. Le Gouvernement, comme l'administration, s'arc-boute sur des schémas du XX siècle, en restant habité par cette mystique qui veut que la grandeur de la France passe nécessairement par une industrie nucléaire triomphante. La puissance du nucléaire, oui, mais avec quelles conséquences ? La construction de nouveaux EPR dans les prochaines décennies est plus qu'aventureuse, au niveau technique aussi bien que financier. Comme le montre l'EPR de Flamanville, l'industrie nucléaire française ne maîtrise pas ce genre de chantiers. Alors qu'il devait être opérationnel en 2012, cet EPR ne le sera pas avant 2023. Et son coût a a été multiplié par six- une bagatelle ! Pour l'instant ! EDF est au bord de la faillite et l'argent public devrait être mieux utilisé. Ces prétendus fleurons de l'industrie française nous coûtent cher, très cher, excessivement cher. Ces réacteurs n'ont aucune chance d'être rentables sur le marché électrique européen. Le choix du nucléaire pose des problèmes majeurs de sûreté, de sécurité et de déchets. Dix ans après la catastrophe de Fukushima, qui a cruellement rappelé à la communauté internationale les dangers de cette industrie, nous ne pouvons plus jouer les apprentis sorciers.

notre vulnérabilité est extrême avec l'industrie atomique. Alors que nos fleuves sont au plus bas en été, la poursuite du nucléaire, c'est un pari fait en regardant dans une boule de cristal. Parlons également de nos vieux réacteurs. L'échelonnement des travaux de remise aux normes pour autoriser la poursuite de l'exploitation au-delà de quarante ans est une prise de risque très importante, surtout au vu de l'accumulation d'incidents graves ces dix dernières années. L'Institut de radioprotection et de Et il n'y a pas que l'argent qui compte ! Sur la question des déchets nucléaires, qu'on ne sait tout simplement pas gérer, dans quelle langue écrire « attention danger » pour des produits dont la durée de vie excède de loin 10 000 ans, quand l'invention de l'écriture date d'environ 5 000 ans ?

Bien sûr, un certain nombre de conditions devront être réunies pour garantir à la fois la sécurité de l'alimentation en électricité, la disponibilité de réserves opérationnelles, la stabilité de la fréquence du système électrique et, enfin, le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution.

Le funeste projet Hercule, négocié dans une opacité totale, est profondément antidémocratique. Il illustre tout ce qu'il ne faut pas faire en la matière. Le nucléaire et la démocratie n'ont décidément jamais fait bon ménage. Pendant ce temps, Photowatt, le seul producteur européen de panneaux photovoltaïques, se meurt. La position des sénateurs et sénatrices écologistes est claire.

je vous remercie Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « la politique publique énergétique de notre pays est marquée du sceau de l'indécision ». C'est ce que l'on peut lire dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution qui nous rassemble aujourd'hui.

Bien au contraire ! Pour conforter notre souveraineté énergétique, il est simplement nécessaire de ne pas dépendre d'une seule source. Il y a le nucléaire, bien sûr, et nous allons y revenir, mais aussi les énergies renouvelables, comme l'éolien, à terre ou sur mer, le solaire, l'hydraulique, la biomasse, la géothermie, entre autres sources. Le code de l'énergie, auquel vous faites référence, vise l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. De telles ambitions sont compatibles avec notre politique énergétique. En effet, ce qui lie toutes ces énergies produites en France, c'est qu'elles sont décarbonées. Nous allons entendre beaucoup de réserves de part et d'autre de cet hémicycle, mais les faits sont là avec une empreinte carbone de 6,9 tonnes par habitant, nous sommes résolument bien placés dans l'Union européenne. L'énergie nucléaire contribue à ce bon classement, elle ne rejette pas, ou très peu, de dioxyde de carbone. Elle produit en moyenne 35 grammes d'équivalent CO2par kilowattheure, contre 1 200 grammes pour les centrales à charbon, charbon qui ne produit que 0,2 % de notre électricité, contre 29 % en Allemagne. Il est à noter la fermeture, en 2022, des quatre dernières centrales à charbon En même temps, nous devons amplifier notre production d'énergies renouvelables. Le projet de loi Énergie-Climat vise un niveau de 33 % de consommation d'énergie d'origine renouvelable en 2030. C'est un objectif atteignable. La part des énergies renouvelables dans la consommation finale a beaucoup progressé ces dernières années. Les EnR ont ainsi participé, à hauteur de 26,9 %, à la couverture de la consommation de notre électricité l'année dernière. Il s'agit d'une progression de près de quatre points par rapport à 2019, mais c'est un chiffre à manier avec prudence au vu de la mise à l'arrêt d'une partie de nos entreprises pour cause de covid. nous sommes capables d'atteindre de bons résultats. Le Gouvernement maintient ce cap et va injecter 30 milliards d'euros pour la transition écologique le plan de relance, 2 milliards d'euros étant dédiés à la filière de l'hydrogène vert, un soutien qui pourrait atteindre 7 milliards d'euros d'ici à 2030, ce qui ferait de la France un pays moteur en la matière. Parlons également de l'éolien en mer, qui tarde à se développer au large de nos côtes. D'ici à 2026, 7 parcs éoliens devraient être construits. Ainsi, plus de 350 éoliennes devraient turbiner dans les eaux françaises. Je souhaite aussi parler du nucléaire. C'est d'ailleurs la principale inquiétude qu'exprime cette proposition de résolution, dont les auteurs estiment « nécessaire de préserver l'atout industriel et technologique que représente cette filière ». Sur ce point, nous sommes d'accord ; nous le sommes d'autant plus qu'à notre connaissance le Gouvernement partage pleinement ce point de vue. Le Président de la République l'a rappelé le 8 décembre dernier au Creusot : « Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Nous assumons cette position, que nous ne sommes pas les seuls à avoir en Europe, puisque d'autres pays, comme la Finlande ou les Pays-Bas, se sont engagés dans cette voie en étudiant la réalisation de nouveaux réacteurs nucléaires. À ce sujet, alors que l'EPR de Flamanville accumule, il est vrai, les déconvenues, un travail d'étude sur la construction de nouveaux réacteurs est en cours pour garantir, en particulier, un niveau de sûreté maximal. En règle générale, nous devons poursuivre nos efforts en matière de gestion des déchets et maintenir notre vigilance sur la capacité de résistance des piscines d'entreposage des combustibles nucléaires usés. Le nucléaire, ce sont aussi, comme le précise cette proposition de résolution, 2 600 entreprises réparties dans les territoires et employant plus de 220 000 salariés. C'est véritablement une ressource économique puissante et un réseau territorial de sous-traitants sans précédent. Le nucléaire, c'est aussi un potentiel d'avenir. Le plan de relance y injectera d'ailleurs 500 millions d'euros, dont 100 millions d'euros dès cette année pour moderniser et transformer ce secteur stratégique. viens d'un département, la Drôme, où l'énergie nucléaire occupe une place importante, tant dans l'économie locale que dans la production française, avec notamment la centrale du Tricastin, Cruas-Meysse étant juste de l'autre côté du Rhône. Ces deux centrales représentent 12 % de la production française. Je mesure donc l'intérêt de cette production. Nous le mesurons d'autant plus que, avec les élus de nos territoires- 175 signataires parmi nos parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, maires et présidents d'EPCI de toutes les sensibilités politiques -, nous avons fait connaître au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy, notre soutien total pour accueillir l'EPR 2 sur le site du Tricastin,

Ces petites unités sont plus faciles à installer et moins complexes à brancher aux réseaux électriques. Avec ces projets, la France vise l'export, mais nous ne devons pas tarder, car nous ne sommes pas seuls sur ce nouveau marché : la Chine, la Russie et les États-Unis sont déjà dans la course. Enfin, l'urgence climatique nous impose d'agir sur notre consommation d'énergie finale. L'exposé des motifs précise que la baisse observée entre 2012 et 2019 est insuffisante. Pour autant, plutôt que de nous focaliser sur le verre à moitié vide, agissons ! C'est ce que fait cette majorité. En témoignent le succès retentissant de MaPrimeRénov'-

pour enrichir notre mix énergétique, et nous y arriverons. Pour ces raisons, rejetant le déclinisme qui irrigue l'ensemble de cette proposition de résolution, le groupe RDPI votera contre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nombreux sont les États, les collectivités territoriales et les entreprises qui se sont engagés sur l'objectif de neutralité carbone en 2050, un défi sans précédent. La Commission européenne propose quant à elle de porter à 55 % l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, soit en moins de dix ans. L'analyse des motifs de la proposition de résolution est pertinente. Elle suppose un basculement important des énergies fossiles vers l'électricité, essentiellement d'origine décarbonée en France, et ce grâce au nucléaire. La stratégie nationale bas-carbone repose sur une augmentation de la part de l'électricité de 25 % à 50 % des besoins énergétiques finaux d'ici à 2050. Les risques de la réduction de la part du nucléaire au sein de notre mix électrique, en ce qui concerne tant la sécurité d'approvisionnement que la stabilité du système électrique, ne peuvent pas être minimisés. La prolongation de la durée de vie des 32 réacteurs de 900 mégawatts de quarante à cinquante ans, décidée en février par l'Autorité de sûreté nucléaire, constitue une bonne nouvelle, mais cela ne suffira pas face à la faible disponibilité du parc nucléaire et à la demande croissante en électricité à venir. Dans ces circonstances, l'abandon progressif du recours au gaz pour le chauffage des logements par la nouvelle réglementation thermique RT 2020 est prématuré. De même, au nom du respect de l'environnement et de la lutte contre la pollution, la puissance publique demande aux Français de remplacer le chauffage au charbon et au fioul par des pompes à chaleur électriques et les incite à remplacer leurs véhicules fonctionnant au diesel par des véhicules électriques ou hybrides ; mais, à terme, l'ensemble de ces décisions aura pour conséquence une augmentation exponentielle de la consommation électrique dans notre pays. Malgré le report de la construction de 6 nouveaux EPR, le soutien apporté à la filière nucléaire par le Président de la République lors du discours du Creusot, en décembre dernier, est sans équivoque : « Notre avenir écologique et énergétique passe par le nucléaire. » Nos collègues s'insurgent contre le rapport commandé par le Gouvernement à RTE et à l'Agence internationale de l'énergie afin d'étudier la faisabilité technique d'un mix électrique avec un très haut niveau d'intégration d'énergies renouvelables. Huit scénarios principaux sont à l'étude, avec une pondération du nucléaire située entre 0 % et et 50 % à l'horizon 2050. Nous considérons que cet exercice de prospective est utile, car il permettra d'anticiper les obstacles techniques, financiers, environnementaux ou sociaux à venir

S'il est vrai qu'il faut veiller à ne pas tomber en situation de pénurie énergétique et qu'il est nécessaire de décarboner notre mix énergétique, d'autres variables, loin d'être négligeables, sont absentes de l'équation établie par la proposition de résolution la montée en puissance des énergies renouvelables, les économies d'énergie et le développement du stockage de l'énergie. Il faut donner un coup d'accélérateur aux énergies renouvelables, devenues désormais compétitives. Paradoxalement, les recours contre les parcs éoliens ou photovoltaïques se multiplient partout. Voilà quelques semaines, dans mon département de une décision de justice a été rendue à la suite de l'action d'une association dite environnementale contre un parc éolien. Ce dernier a été condamné à la destruction.

Le stockage de l'énergie doit aussi évoluer. Je pense à l'hydrogène vert, comme je l'ai souligné le 18 novembre dernier, lors du débat mis à l'ordre du jour du Sénat à la demande du groupe RDSE sur le thème : « La France peut-elle devenir un champion de l'énergie hydrogène ? » l'avenir, il convient, à mon sens, de conserver notre parc nucléaire tant que d'autres solutions ne nous permettront pas de répondre aux besoins du pays en toute indépendance énergétique. même temps, il faut développer les énergies renouvelables et rénover notre parc de logements, avec une volonté forte et des financements importants de la part de l'État. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution sur la mise en cohérence de la politique énergétique du Gouvernement avec ses ambitions environnementales est essentiellement axée sur la place de la production électrique d'origine nucléaire dans notre mix énergétique. Je souhaite l'aborder sans dogmatiques, loin des positions « anti-énergies renouvelables » ou « anti-nucléaire qui ne permettent pas, selon nous, un débat serein, et empêchent de saisir les véritables enjeux auxquels nous sommes confrontés aux échelles nationale et mondiale : l'urgence d'une révolution environnementale globale ; l'exigence de sortir 12 millions de nos concitoyens de la précarité énergétique ; la sécurisation et la garantie pour les décennies futures de notre souveraineté énergétique. La question est celle de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour l'atteindre, comment bâtir une meilleure complémentarité entre les différentes énergies ? L'évolution de notre système électrique impliquera la construction de nouveaux moyens de production, le développement de nouvelles filières industrielles et de nouvelles infrastructures de réseau. Cela suppose non seulement de planifier et mobiliser des moyens financiers qui s'inscrivent sur le temps long, mais aussi de continuer à investir dans la recherche et le développement. C'est pourquoi il est impératif de sortir des confrontations entre positions tranchées pour que les choix technologiques ne soient plus l'apanage de l'exécutif, en particulier du Président de la République, mais qu'ils résultent bien d'un choix citoyen éclairé. Le nucléaire est aujourd'hui un atout incontestable. Nous sommes d'accord ! Il s'agit de l'énergie la plus décarbonée, qui permet une maîtrise des coûts, même si les importations d'uranium ne sont pas prises en compte dans la facture énergétique française. C'est surtout une énergie pilotable, contrairement aux énergies renouvelables aujourd'hui, ... Oui ! ... et donc un atout pour éviter le blackout. Le fait de renoncer aux centrales à charbon va renforcer cette dépendance au tout-nucléaire. Toutefois, nous ne pouvons occulter l'impact majeur des accidents de Tchernobyl et Fukushima sur l'acceptation par nombre de nos concitoyens de notre dépendance à ce mode de production.

Pourtant, rien n'est dit sur l'échec de la libéralisation de l'électricité ni sur l'Arenh, qui oblige EDF à vendre une partie de sa production nucléaire à ses concurrents. Exact ! Or, mes chers collègues, je suis désolé de vous le dire, mais ce bilan est le vôtre. Il a provoqué des augmentations de tarifs pour les usagers. Pire, l'Autorité de la concurrence nous rappelle que 40 % des augmentations des tarifs réglementés « ont pour but de permettre aux concurrents d'EDF de proposer des prix égaux ou inférieurs à ces tarifs ». C'est donc aux ménages de supporter la note en payant le prix de l'Europe libérale au profit des actionnaires des opérateurs alternatifs. Pourtant, ces tarifs réglementés sont la garantie pour chacun d'avoir accès à l'énergie et l'un des atouts pour la compétitivité de nos entreprises. Enfin, vous nous dites qu'il ne faut pas « fragiliser davantage l'opérateur historique de production d'électricité et ses salariés ». En ce cas, pourquoi ne pas demander clairement au Gouvernement de renoncer au projet Hercule, hérité du dogme dépassé des bienfaits de la concurrence libre et non faussée ? Nous savons tous ici qu'il ne vise qu'à créer de la concurrence là où il ne peut y en avoir. Vous le savez, si ce projet est adopté, alors, la filière nucléaire, qui sera 100 % nationalisée dans « EDF Bleu » sera lourdement handicapée en raison de la séparation avec les autres activités, qui seront ainsi privatisées. On fera peser la dette sur cette structure EDF Bleu, alors que le nucléaire a besoin dans les années à venir des plus grands investissements pour sécuriser et démanteler les centrales qui devront l'être, pour se développer. Pour nous, la complémentarité entre énergies doit se faire dans un groupe qui reste intégré et dispose d'un monopole public. Pour conclure, je dirai que l'intérêt général, l'environnement et l'accès à l'énergie pour tous

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe Les Républicains d'avoir déposé cette proposition de résolution. Je crois déterminant pour les parlementaires de discuter de la politique énergétique du Gouvernement, car le court terme de la crise sanitaire ne doit pas faire oublier le défi sur le long terme du dérèglement climatique. Si l'exécutif en a conscience, comme en témoigne le projet de loi Climat et résilience, comment expliquer le nombre dérisoire de dispositions dans ce texte se rapportant à l'énergie ? La question n'est abordée quasiment que sous le prisme de la rénovation énergétique. Certes, l'enjeu est important, mais cela ne suffira pas pour atteindre les objectifs affichés La réduction massive de nos émissions de gaz à effet de serre doit passer par la production d'une énergie décarbonée. Or, sur ce sujet, le projet de loi fait montre d'une frilosité que je déplore. En parallèle, une étude de RTE est venue affirmer la faisabilité d'un scénario « 100 % énergies renouvelables » d'ici à 2050. Si je doute que le projet soit techniquement et administrativement réalisable, il ne me paraît pas non plus souhaitable. En effet, les EnR, telles que le photovoltaïque ou l'éolien, sont par nature intermittentes, non pilotables, et l'électricité qu'elles produisent n'est pas stockable en l'état actuel de la technologie. Ces limites ont pris un caractère très concret quand RTE a demandé en janvier à nos concitoyens de réduire leur consommation électrique pour éviter des coupures localisées sur le réseau. ont ainsi pu constater les difficultés des éoliennes à prendre le relais du parc nucléaire quand le vent vient à manquer. De plus, de nombreux projets d'EnR sont contestés par les citoyens et les associations environnementales. Alors, effectivement, d'autres énergies renouvelables ont des atouts à faire valoir, avec des emplois non délocalisables et une exploitation valorisant nos territoires, territoires, surtout ruraux. Je pense, par exemple, au biogaz issu de la méthanisation agricole, qui peut aisément être injecté dans les réseaux de gaz naturel et s'y substituer. Cependant, le Gouvernement semble réticent à lui témoigner sa confiance la RE 2020 qu'il souhaite faire appliquer conduirait, dans les faits, à écarter son usage pour chauffer les bâtiments neufs. Quant aux barrages hydroélectriques, leur sort est toujours suspendu aux résultats des discussions avec la Commission européenne, ce qui bloque des investissements pourtant nécessaires pour moderniser les infrastructures. Enfin, le développement de l'hydrogène paraît prometteur, mais la filière doit encore se structurer pour être à la fois rentable et écologique, ce qui va prendre du temps. Dans ces conditions, je pense, comme le Président de la République, que le nucléaire doit faire partie de la solution, car c'est une énergie décarbonée. Malheureusement, le sort de la filière semble aujourd'hui lié au dangereux projet C'est pourquoi je souhaite que le Gouvernement clarifie sa position en la matière dès que possible pour redonner des perspectives à celle-ci. En parallèle, l'industrie nucléaire doit encore convaincre les Français à la fois sur sa sécurité et sur son coût. Il lui reste beaucoup à prouver, alors que la mise en service de l'EPR de Flamanville risque d'être de nouveau retardée et que les centrales existantes doivent être aménagées pour que leur fonctionnement Le nucléaire doit évidemment faire partie de notre politique énergétique si nous voulons être à la hauteur de nos ambitions écologiques. Il ne doit pas pour autant en constituer l'unique horizon. Union Centriste votera majoritairement ce texte. Quant à moi, je m'abstiendrai eu égard aux arguments que je viens de développer devant vous.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour, je remercie les auteurs de cette proposition de résolution, qui nous permet aujourd'hui de débattre des enjeux très importants que représente notre avenir énergétique. représente notre avenir énergétique. Ce texte invite le Gouvernement « à étudier la possibilité d'une mise en cohérence de sa politique énergétique avec ses ambitions écologiques ». Ce titre est encourageant, car il met sur un pied d'égalité la politique énergétique, la cohérence et les ambitions écologiques.

L'impossibilité de contrôler notre consommation énergétique, exprimée par ses auteurs, est un premier point important de divergence. Il n'est pas irréaliste d'imaginer une consommation énergétique plus sobre et respectueuse de notre environnement et de nos ressources. Seule une réelle volonté politique permettra d'atteindre cet objectif. Le deuxième point de divergence est le tout-nucléaire prôné par les auteurs de la proposition de résolution. Pour l'avenir de la politique énergétique de notre pays, nous ne devons pas nous laisser enfermer dans une opposition stérile entre les pro-nucléaires et les anti-nucléaires. Les réalités structurelles, techniques et matérielles du secteur de l'énergie doivent nous conduire à trouver un juste milieu. Non, nous ne pourrons pas nous passer de l'électricité d'origine nucléaire du jour au lendemain. Oui, les énergies renouvelables occupent une place croissante dans notre bouquet énergétique, grâce à des innovations régulières et une mobilisation de plus en plus importante. Face à ces enjeux, le Gouvernement fait preuve d'une impréparation et d'une inaction inquiétantes. En début d'année, le débat sur le risque de blackout énergétique nous avait permis d'exprimer nos opinions respectives sur la stratégie énergétique de notre pays. Nous avions notamment souligné les retards pris pour l'entretien des centrales nucléaires. Alors que nous sortons juste de l'hiver 2021, l'utilisation à vingt-deux reprises de la centrale à charbon de Saint-Avold et l'importation d'électricité d'origine allemande, produite à 40 % par des ressources fossiles, sonnent comme des échecs pour la décarbonation de notre énergie. Afin de mettre en cohérence la politique énergétique de notre pays avec les ambitions environnementales fixées par les accords de Paris, seule une véritable planification de la transition écologique permettra de programmer sur le long terme la décarbonation de nos modes de production et la transformation de nos modes de consommation. Notre politique énergétique doit s'inscrire dans une vision où seraient réellement planifiés la rénovation thermique des bâtiments, le développement des mobilités propres et un plan d'investissement pour la reconversion industrielle, avec des mesures d'accompagnement social pour les secteurs impactés. Le rééquilibrage de notre bouquet énergétique, engagé lors de la mandature précédente par la ministre de l'environnement, Ségolène Royal, s'inscrit aussi dans cette programmation. La réduction progressive de la part du nucléaire au profit des énergies renouvelables doit se poursuivre à l'échéance de 2035. La construction de l'EPR de Flamanville sonne elle aussi comme un véritable échec avec ses multiples retards et ses surcoûts. Elle révèle la défaillance de l'État actionnaire, qui préfère optimiser ses participations financières au détriment du pilotage sur le long terme de l'outil industriel. En matière d'énergies renouvelables, les estimations réalisées par RTE sont encourageantes : les EnR ont participé à près de 30 % de la consommation d'électricité en France métropolitaine en 2020. L'éolien est même devenu la troisième source de production d'électricité. Ce contexte implique pour le Gouvernement et la représentation nationale de disposer d'une vraie capacité à mettre en oeuvre une politique énergétique maîtrisée et souveraine. Pourtant, en se désengageant progressivement de certains grands groupes du secteur de l'énergie,

L'esprit libéral de ce gouvernement va malheureusement à l'encontre des enjeux et des nécessités de notre époque. La question d'un véritable service public de l'énergie mérite d'être posée et ne doit pas être balayée d'un revers de main. Sur un secteur aussi stratégique, les les décisions que nous prenons aujourd'hui se répercuteront sur les générations de demain. Ainsi, mes chers collègues, pour souligner combien les enjeux relatifs aux changements climatiques supposent d'agir simultanément sur nos modes de production et de consommation de masse, énormément consommateurs d'énergie, le groupe Socialiste,

À défaut de l'avoir obtenu, je me réjouis que la présente proposition de résolution l'ait provoqué. Au printemps dernier, la pandémie de la covid-19 a plongé le secteur de l'énergie dans une crise tout à fait inédite, après une chute de 5 % de la demande mondiale. C'est pourquoi l'Agence internationale de l'énergie estime que la crise sanitaire a causé plus de perturbations que tout autre événement dans l'histoire récente. Dans ce contexte, les projets de restructuration se multiplient, Après le projet Hercule et le projet Bright, même TotalEnergies revoit certains de ses objectifs. Cette succession d'annonces, globalement pose de lourdes questions pour notre souveraineté et notre transition énergétiques. Concernant notre souveraineté, nous assistons à un long affaiblissement de notre appareil

De son côté, Engie restructure les deux tiers de ses activités de services, avec des répercussions sur la moitié de son personnel. Que dire enfin de la cession, il y a quelques années, des turbines nucléaires d'Alstom à General Electric ? La situation nous semble préoccupante. Face à ces difficultés, notre commission n'a pas ménagé ses efforts. Tout d'abord, elle a reculé de dix ans l'objectif de réduction à 50 % de la proportion d'énergie nucléaire dans le cadre de la loi Énergie-climat. Sans cela, le nombre de fermetures de réacteurs aurait atteint dès 2025 ! Étions-nous prêts à faire face ? Eh bien, je vous le dis : nous n'étions pas prêts. Par ailleurs, notre commission poursuit une intense activité de contrôle, notamment sur EDF et Engie. Si notre souveraineté est ainsi mise à l'épreuve, il en va de même de notre transition vers une économie plus sobre en carbone. La recherche nucléaire semble en berne depuis l'arrêt du réacteur Astrid ; les énergies renouvelables ne sont pas mieux loties, avec la remise en cause de dispositifs de soutien

l'énergie est en réalité issue de redéploiements de crédits. De toute évidence, ces moyens sont bien insuffisants pour relancer notre économie en accélérant sa décarbonation. Dès le mois de juin dernier, notre commission avait pourtant proposé d'investir massivement dans l'industrie nucléaire, la rénovation énergétique et les énergies alternatives. Je ne vois aucune opposition entre le développement du nucléaire et les efforts sur les autres points énergétiques. Aujourd'hui, nous attendons du Gouvernement qu'il sorte d'un double déni : il doit admettre que la crise de la covid-19 a un impact considérable sur le secteur de l'énergie, mais aussi que nous devons faire davantage

Face à l'urgence climatique, il faut cesser de tergiverser sur les avantages et les inconvénients du nucléaire, car nous n'accomplirons pas la transition actuelle vers une économie sobre en carbone sans le nucléaire : celui-ci est le meilleur allié l'évolution du climat (GIEC) qui le dit. Alors il nous faut accélérer l'achèvement de l'EPR de Flamanville, cher Daniel Gremillet ; il nous faut développer les trois paires d'EPR ; il nous faut dynamiser les projets du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et, bien sûr, conforter les missions de l'Autorité de sûreté nucléaire, missions qui sont tout à fait essentielles pour la confiance des Français. L'hydrogène nucléaire doit aussi être activement soutenu, à l'échelle nationale comme au niveau européen, car il permet le développement de la filière aval en attendant l'hydrogène vert. Voilà, monsieur le ministre, ce que nous attendons du Gouvernement. C'est plus substantiel et, peut-être, plus ambitieux que certaines dispositions du projet de loi Climat et résilience, dont on peut s'étonner qu'il soit absolument muet sur l'énergie nucléaire. Je forme donc le voeu que celle-ci retrouve une place de choix dans notre mix énergétique, ainsi que dans notre recherche et développement. Cette place n'évincerait en rien le développement légitime et nécessaire des énergies renouvelables.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution déposée par nos collègues du groupe Les Républicains pose la question de l'équilibre à trouver entre la politique énergétique de notre pays et ses ambitions écologiques. Au coeur de ce questionnement figurent nos choix en matière d'énergie nucléaire- avenir des réacteurs de quatrième génération, prolongement ou fermeture des réacteurs actuels -, ainsi qu'en matière d'énergies renouvelables. Pour ma part, il me semble que l'équation que nous avons à résoudre réside plus dans la balance à trouver entre le prix de l'énergie produite et consommée, d'une part, et le mix énergétique que nous souhaitons mettre en place à l'avenir dans notre pays, d'autre part. Même si notre volonté commune est de diminuer nos consommations énergétiques,

relevées dans de nombreuses activités, comme le télétravail ou les usages numériques, impliqueront irrémédiablement une augmentation globale des besoins en énergie électrique. Nous devons donc trouver des sources d'énergie qui assureront l'approvisionnement du pays pour les habitants comme pour les entreprises. Pour cela, il nous faudra être très vigilants quant à notre capacité à produire suffisamment et de manière responsable, au bon moment et surtout au bon prix.

aussi de développer les énergies renouvelables, par l'intermédiaire de l'éolien, du solaire, des biocarburants et, bien sûr, de l'hydroélectrique, dont nous aurons l'occasion de parler prochainement. produire au bon moment. C'est à l'évidence une autre des qualités du nucléaire, mais cela doit aussi nous inciter à accentuer la recherche et développement en matière de stockage de l'électricité. enfin, produire au bon prix : c'est sans doute la plus grande difficulté. L'Arenh a déjà permis de favoriser l'émergence de fournisseurs d'électricité alternatifs, sans leur faire porter la charge de l'investissement et de la recherche sur le nucléaire. Le projet Hercule, demandé à EDF par le Gouvernement, possède comme principal ressort l'évolution de cet accès régulé. Ce boulet aux pieds de l'opérateur historique ne lui permet ni d'amortir ses coûts ni d'investir pour l'avenir dans le nucléaire et les énergies renouvelables. Où en sont, monsieur le ministre, les négociations avec la Commission européenne sur cette question primordiale pour EDF, pour l'organisation du secteur énergétique en France et pour les consommateurs français ?

l'on souhaite passer de 70 % à 50 % de nucléaire dans le mix à l'horizon 2035, prenons garde à nous doter de la capacité d'investir dans d'autres sources d'énergie décarbonées suffisamment productrices Il serait incompréhensible de devoir importer de l'électricité parfois produite à partir de charbon. L'Europe possède le plus grand parc nucléaire du monde ; il représente en fin de compte une partie de la solution pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050. Néanmoins, les dynamiques mondiales démontrent que ce sont la Chine et la Russie qui ont les dynamiques de capacités de mise en service les plus importantes, la Chine devant dépasser l'Europe vers 2030. L'Europe est donc à la croisée des chemins. Au-delà d'une question purement nationale, nous devons élever le débat et impulser une véritable politique européenne de l'énergie, qui soit ambitieuse, décarbonée et indépendante. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, oui, nous devons mettre en cohérence la politique énergétique de la France avec ses ambitions écologiques. dit, notre production d'électricité est aujourd'hui fortement décarbonée, à 93 %, dont plus de 70 % de nucléaire. La part des énergies renouvelables dans notre production augmente régulièrement, mais il faudrait s'engager de manière plus volontariste encore dans leur développement pour compenser les futures fermetures de centrales, sans oublier l'hydroélectricité, qui est tout de même la seule énergie renouvelable capable d'assurer le maintien des réseaux et des fréquences ; la petite hydroélectricité, très pertinente à l'échelon local, est pourtant sujette à de nombreux freins. En réalité, pour décarboner, l'impératif est de réduire la consommation d'énergie fossile dans les secteurs les plus émetteurs c'est-à-dire en premier lieu dans les transports. Une révolution de nos mobilités et de nos modes de consommation et de production est donc incontournable et nécessaire. Une réflexion doit également être menée sur les déchets et le gaspillage. conditionner les aides publiques en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone et d'investir davantage dans le financement de la transition écologique : 50 milliards d'euros de plus par an sont nécessaires,

de travaux dans le cadre du « grand carénage ». S'ajoute à cela le fait que le réchauffement climatique s'installe de manière pérenne sur nos territoires : l'augmentation de la température des fleuves et la trop grande faiblesse des débits ne permettent plus d'assurer le refroidissement, entraînant des arrêts répétés de certaines centrales. C'est le cas de celle refroidie par la Garonne, qui atteint 30 degrés tous les étés, vrai sujet d'inquiétude. Il faut ensuite se pencher sur le fiasco technologique et économique de l'EPR de Flamanville, qui devait être raccordé au réseau en 2012 et coûter 3,3 milliards d'euros. Or on a appris le 16 mars dernier qu'il y avait encore des problèmes de soudure ; l'ASN a demandé à EDF de lui indiquer sa stratégie et les raisons de la détection tardive de ces problèmes. Au mieux, cette centrale sera raccordée au réseau en 2023 et devrait coûter quatre à six fois plus cher que prévu. Dès lors, comment envisager l'avenir du nucléaire ?

comme définitivement acquise ». Un accident nucléaire en France, ce serait un demi-département rayé de la carte, qu'on ne pourrait même plus traverser, contaminé pour des milliers d'années ; ce serait des centaines de milliers de personnes déplacées et une centrale qu'il faudrait refroidir sans cesse. À Fukushima, en ce moment, on injecte en continu de l'eau douce dans les cuves des réacteurs 1, 2 et 3. Quant à l'exploitation minière de l'uranium, elle n'a pas toujours été des plus vertueuses, en France comme ailleurs.

porte sur un sujet sociétal par excellence, il serait absolument nécessaire d'y associer nos concitoyens : après tout, on ne leur a jamais demandé leur avis sur cette question, choix crucial d'avenir mêlant souveraineté, indépendance, industrie et écologie. Pour une fois, il serait bon de bien faire les choses, c'est-à-dire de donner à nos concitoyens des connaissances pour leur offrir les conditions d'un choix éclairé. Pour toutes ces raisons, la diminution de la part du nucléaire actée dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, jusqu'à 50 % en 2035, nous paraît un choix raisonnable. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur cette proposition de résolution. La parole

Dans son rapport de mars 2020, la Cour des comptes indique que la fermeture de Fessenheim se caractérise par un processus de décision chaotique. De fait, cette fermeture est une triple faute. tout d'abord une faute écologique et l'amorce d'un écocide. Les deux réacteurs de Fessenheim représentaient une production de 1,8 gigawatt. Avec la centrale de Fessenheim, RTE n'aurait pas été obligé de tirer la sonnette d'alarme cet hiver : nous n'aurions pas eu de tensions sur les réseaux.

Par conséquent, si votre délit d'écocide est correctement appliqué, les personnes qui ont décidé de la fermeture de Fessenheim pourraient être poursuivies, puisque cette décision a été néfaste pour l'environnement de la centrale de Fessenheim est une faute économique et industrielle. Comme le dit le maire de Fessenheim, la centrale était un îlot de prospérité. La fermer a mis en difficulté 2 000 emplois directs et indirects, ainsi que les familles

Fermer Fessenheim a aussi eu des conséquences pour nos finances publiques. On a dû verser 400 millions d'euros à EDF pour sa fermeture, sans compter toutes les sommes à ajouter pour le manque à gagner ; le coût du démantèlement est évalué à 2 milliards d'euros. Alors, monsieur le ministre, pourquoi fermer Fessenheim ? Était-ce parce que la centrale était la doyenne du parc, ou qu'elle était trop vieille ? L'âge d'une centrale n'a rien à voir avec sa sûreté ; c'est d'ailleurs ce qu'indiquent les différents rapports. La centrale était sûre et rentable ; elle pouvait encore fonctionner durant plusieurs années, comme l'indique l'Autorité de sûreté nucléaire. C'est là qu'intervient la troisième faute, qui laissera des traces sur notre territoire

Ils n'oublieront pas que Fessenheim a été sacrifiée pour quelques voix et un accord électoraliste entre le PS et les Verts en 2012. Sacrifier des intérêts stratégiques et économiques, un territoire et les salariés sur l'autel d'un accord politicien, c'est une erreur historique ! Enfin, la reconversion du territoire n'a pas été anticipée et le projet de technocentre, une usine de traitement de métaux radioactifs, est très loin des attentes. Ce projet, défendu par le Gouvernement, verrait une mise en service au plus tôt en 2029 avec seulement 150 emplois créés : on aura vu mieux comme reconversion

Après la fermeture des réacteurs de Fessenheim et la fin de non-recevoir sur StocaMine, l'attente est forte sur le territoire alsacien. Pour l'instant, monsieur le Nous devons, collectivement, assurer cette reconversion du territoire. Les élus sont prêts à vous suivre, mais sur un projet viable. Avec le plan de relance, nous avons une chance inouïe d'assurer cette reconversion : il prévoit 200 millions d'euros pour la filière nucléaire. Alors fléchons dès aujourd'hui une partie de ce fonds pour la reconversion du territoire de Fessenheim ! La parole

pour votre invitation, qui me permet de vous exposer la cohérence de notre politique énergétique avec nos ambitions écologiques. Cette cohérence s'apprécie déjà dans nos objectifs, nos ambitions et nos investissements. Ce qui nous fait défaut, en matière d'énergie, ce n'est pas tant la cohérence que la souveraineté. Le grand défi de notre génération et des suivantes, après presque deux siècles d'abondance énergétique, est de garantir notre sécurité d'approvisionnement dans des conditions soutenables pour la planète. faire, nous devons donner à la France les moyens de sa souveraineté énergétique. En matière d'énergie comme pour les autres secteurs stratégiques, la souveraineté repose sur la diversification et l'indépendance. Cette stratégie est un héritage : nous le devons au Conseil national de la Résistance, qui donna naissance à EDF et GDF, deux sociétés d'impulsion étatique qui constituent depuis lors des attributs de puissance de la France et ont été un moyen pour le pays de se reconstruire, mais aussi l'un des fondements de son identité. le gaz, nous avons constitué au fil des années l'un des portefeuilles d'approvisionnement les plus diversifiés d'Europe. C'est une force ; tous nos voisins ne peuvent pas en dire de même. Pour l'électricité, avec le développement du nucléaire, comme cela a été rappelé, nous avons construit un atout précieux : celui d'avoir une électricité parmi les moins carbonées au monde. Comme vous le savez, nous avons fait le choix de ramener progressivement la part du nucléaire de 70 % à 50 % du mix électrique d'ici à 2035. Viser 50 %, c'est maintenir la part prépondérante du nucléaire en France et c'est préserver une filière de 2 600 entreprises et de plus de 200 000 emplois directs et indirects ; ces chiffres aussi ont été cités dans ce débat. Il nous revient aujourd'hui de terminer les grands chantiers actuels et de préparer ceux qui s'annoncent. Il s'agira aussi de constituer une filière de démantèlement et de développer de nouvelles solutions pour le traitement des déchets. Pour cela, la filière nucléaire peut compter sur un savoir-faire et une excellence reconnus à travers le monde. Mais elle doit aussi pouvoir compter sur une capacité d'investissement que le Gouvernement renforce avec France Relance. Nous mobilisons ainsi un demi-milliard d'euros pour soutenir les entreprises les plus sensibles, pour amplifier l'effort de recherche et développement, pour renforcer les compétences critiques et pour moderniser une industrie qui fait l'honneur de la France depuis soixante Parallèlement, nous devons accélérer le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, celles-ci fournissent déjà environ un cinquième de notre production électrique, notamment parce que nous avons historiquement développé l'hydraulique. Ces énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives. Nous pouvons passer à la vitesse supérieure, avec un cap clair : que, d'ici à 2030, 40 % de l'électricité produite dans le pays soit renouvelable. Pour cela, nous devons développer plus largement le solaire, l'éolien et l'hydrolien. Concernant le solaire, nous avons pour objectif de quadrupler la puissance installée d'ici à 2028, tout en développant des panneaux tant sur les toitures que par des centrales au sol. Quant à l'éolien terrestre, nous devons poursuivre et amplifier nos efforts, tout en nous assurant de l'acceptabilité des projets. L'objectif est de doubler la puissance d'ici à 2028. ou hydrolien, nous avons le deuxième gisement d'Europe par son potentiel. Celui-ci doit être davantage exploité ; la simplification administrative peut nous y aider. Nous avons déjà engagé ce travail dans la loi ASAP, mais nous pouvons faire davantage. Par ailleurs, un certain nombre d'études montrent que nous pourrions intégrer des taux supérieurs à 40 % d'énergies renouvelables variables sans mettre en péril la sécurité du système électrique. Comme vous le savez, RTE analyse actuellement des scénarios de long terme. Ces travaux nous seront remis à l'automne seront- je n'en doute pas -de nature à nourrir le débat et à éclairer les décisions qui seront prises au début du prochain quinquennat. Mais notre mix énergétique ne se résume pas à l'électricité : il y a aussi le gaz. Pour décarboner cette filière, la solution est non pas de la démanteler, mais bien de la transformer et de développer, pour ce faire, le gaz renouvelable. Nous avons pris des engagements inédits à cet effet dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. En trois ans, nous avons multiplié par quatre le nombre d'installations de méthanisation, qui constituent aussi de plus en plus souvent, comme vous le savez, des compléments de rémunération pour nos agriculteurs. Nos capacités de production augmentent rapidement. Au total, nous investirons 10 milliards d'euros dans le biogaz d'ici à 2028. Enfin, nous devons bâtir une filière française de l'hydrogène qui nous permettra de décarboner un certain nombre d'usages dans les champs de l'industrie et des transports. Pour construire cette filière, il faudra s'assurer de la production d'un hydrogène vert ou décarboné. Pour cela, l'option la moins coûteuse et la plus efficiente est de le produire localement, par électrolyse, à partir de l'électricité de notre réseau, qui, je le disais, présente l'avantage d'être très peu carbonée. Sincèrement, sur ce sujet, nous avons toutes les capacités pour nous imposer comme l'un des leaders mondiaux de l'hydrogène, raison pour laquelle nous investirons 7 milliards d'euros d'ici à 2030. Notre souveraineté énergétique dépend bien sûr de notre mix, mais aussi de notre consommation. En la matière, nous devons aller vers plus de sobriété, par l'innovation technologique et par l'efficacité énergétique. L'objectif est de faire baisser notre consommation finale d'énergie de moitié d'ici à 2050. Les politiques conquérantes de décarbonation des transports et de rénovation thermique des bâtiments y contribueront fortement. Mesdames, messieurs les sénateurs, les décisions en matière d'énergie dépassent très largement l'horizon de nos mandats politiques. Elles engagent les générations à venir et nécessitent de la réflexion, du débat et de la planification. La place de la France dans le monde, sa souveraineté, sa puissance sont intrinsèquement liées à sa production d'énergie. Le général de Gaulle l'avait bien compris ; il visait en la matière l'indépendance et l'excellence. Cette volonté, cette vision, nous en sommes les héritiers. Soyez assurés qu'elle guide, chaque jour, chacune de nos décisions. Notre politique énergétique n'est pas seulement cohérente avec nos ambitions écologiques ; elle est cohérente avec nos ambitions tout court. Et Hercule

Je dis « nouveau », parce que le 18 novembre 2020, déjà, nous débattions sur l'initiative de nos collègues du groupe RDSE sur le thème de l'« Agence nationale de la cohésion des territoires, un an après sa création

Sous une forme ou une autre, il ne se passe pas une semaine de contrôle passée sans que l'aménagement du territoire figure à l'ordre du jour. Aussi, pourquoi parler de nouveau d'aménagement du territoire ? Dans le cas présent, j'ai la faiblesse de penser que la constance avec laquelle le Sénat traite de cette question n'est pas uniquement le fait de ses attributions constitutionnelles. J'ai même la conviction que l'aménagement du territoire, évoqué avec d'autant plus de vigueur que sa réalité, comme politique publique, nous fait profondément défaut. Vous l'aurez compris, la fonction de ce débat est non pas de produire une analyse critique de la politique publique d'aménagement du territoire du Gouvernement, mais bien davantage de lui demander quelle est cette politique.

notre pays a appuyé toutes ses politiques sectorielles sur l'aménagement du territoire. Comme le précisait Michel Debré : « Il faut répondre à ce devoir d'État qui, en termes administratifs, se nomme aménagement du territoire. Comme chacun ici a pu le constater, cette politique publique s'est lentement érodée avec le temps. Nous avons cru d'abord que la décentralisation était un palliatif suffisant à cet abandon : c'était se tromper. Nous avons cru ensuite que le Fonds européen de développement régional (Feder) allait lui aussi se substituer à ce renoncement c'était, là encore, se tromper. Nous avons cru enfin que les métropoles nous conduiraient dans une nouvelle ère, rendant le concept même d'aménagement du territoire inopérant : c'était, une fois de plus, se tromper Manifestement, plusieurs raisons peuvent être avancées pour justifier la disparition de cette politique publique : pour les libéraux, l'aménagement du territoire, c'est la planification, l'amorce du socialisme ; pour les Girondins, c'est une création jacobine ; pour les autres, c'est une discipline placée sous le sceau de l'arbitraire, du clientélisme. je rejette ces trois assertions. La hausse de la dépense publique nous a conduits à sacrifier nos dépenses d'investissement, nous privant ainsi des moyens indispensables à cette politique. À ce stade, j'ose formuler une question savons-nous encore faire de l'aménagement du territoire, en termes d'ingénierie, bien sûr, mais surtout en termes de réflexion, de vision ? Certes, nous avons multiplié les différents plans et schémas

Là encore, je me demande naïvement si cette avalanche de plans n'est pas un palliatif ... Toutes les actions engagées depuis trente ans n'ont pas permis de faire disparaître le sentiment d'éloignement ou de délaissement, à la ville comme dans nos campagnes. C'est même l'effet inverse qui s'est produit Le voeu pieux de l'article 1 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, aux termes duquel « La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations », semble lui aussi bien lointain. De fait, nous nous sommes accrochés trop longtemps au fait métropolitain et à sa théorie du ruissellement, comme nous avons cru que le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication allait redonner à tous les territoires une nouvelle vocation économique. C'est vrai, mais seulement en partie : plus l'économie se digitalise, plus elle se concentre géographiquement. Plusieurs explications méritent d'être nuancées. D'une part, la moitié des étudiants de France se concentre dans les quinze métropoles que comptait le pays au 1 janvier 2017, alors que celles-ci n'accueillent que 27 % de la population française. D'autre part, la fracture numérique est loin d'être comblée puisque, dans les unités urbaines de moins de 100 000 habitants et dans les communes rurales, seuls 60 % des habitants disent profiter des possibilités ouvertes par les nouvelles technologies, contre plus de 80 % dans l'agglomération parisienne. Face à ces difficultés, maintes fois énoncées par le Sénat, les gouvernements ont répondu, non par l'aménagement du territoire, mais avec des politiques éparses de soutien aux territoires en difficulté, qui ressemblent davantage à des soins curatifs, sans garantie de guérison. Pire encore,

En définitive, que devient l'aménagement du territoire ? Il repose sur le volontarisme des collectivités locales, qui, malgré l'instabilité institutionnelle dans laquelle elles évoluent, se substituent désormais à un État omniprésent et omnipotent. Pour cette raison, nous voulons enfin parler de différenciation, pour que chaque territoire puisse se développer comme il l'entend, fort de son histoire, de sa culture, de son patrimoine et de la volonté des femmes et des hommes qui le font vivre.

Ce sont des signaux positifs, qui n'expriment cependant pas une vision stratégique. L'enjeu, aujourd'hui, est de donner une perspective à nos concitoyens, sans opposer l'urbain et le rural- nous devrions d'ailleurs utiliser le couple ville-campagne pour dessiner notre avenir.

La matière ne manque pas pour alimenter les réflexions de l'exécutif. Faut-il être aveugle et sourd pour ne pas comprendre l'aspiration profonde de nos concitoyens, exacerbée par la crise des gilets jaunes, qui a débouché sur un grand débat national, non suivi d'effets ? Faut-il être enfermé à l'Élysée pour ne pas mesurer les effets durables de la pandémie, qui accentuent la migration vers les campagnes : l'exode urbain, après l'exode rural ? Suffit-il d'évoquer l'objectif de zéro artificialisation dans le projet de loi Climat, qui stigmatise les territoires en développement pour régler la question climatique ? Aucune métropole, y compris Paris, ne s'est construite. Le sujet du développement durable concerne tous les territoires. Ces derniers sont la solution aux questions posées par le projet de loi Climat sur le travail, les déplacements, la production et la consommation.

Vous avez l'ardente obligation de préserver, de protéger ce bien commun, que l'on vive dans une petite commune à la campagne ou dans un quartier prioritaire de la

les transports, le logement et l'urbanisme, mais aussi la santé, le numérique, la jeunesse et l'accès aux services publics. Il y a donc non pas « une » mais « des » politiques d'aménagement du territoire. Pour autant- et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'emploi du singulier -, toutes ces politiques ont un même objectif : tenir la promesse républicaine d'égalité, compenser les handicaps territoriaux pour permettre à chacune et à chacun de s'épanouir dans sa vie personnelle, familiale ou professionnelle, quel que soit son lieu de résidence. Nous devons veiller à ce que chaque territoire dispose des moyens de surmonter ses fragilités et de développer son potentiel en fonction de ses spécificités.

Désormais, et pour la première fois, il existe un secrétariat d'État dédié à la ruralité, auprès de la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Mon rôle est d'assurer le suivi et la mise en oeuvre de l'« agenda rural », ce grand plan national en faveur de la ruralité, qui comprend 181 mesures. Les choses avancent bien : à ce jour, 60 % des mesures ont été réalisées et 25 % sont en cours de réalisation. L'agenda ayant été lancé il y a seulement dix-huit mois, il nous reste encore une année pour achever sa mise en oeuvre- soyez assurés que j'y veillerai personnellement

Je peux aussi citer la fracture numérique, pour laquelle oeuvre Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. La généralisation de la 4G, la résorption progressive des zones blanches et l'accélération du déploiement de la fibre sont des grands succès de notre politique d'aménagement du territoire.

L'aménagement du territoire, c'est aussi la politique de la ville, dont est chargée ma collègue Nadia Hai. Nous oeuvrons en faveur des quartiers défavorisés une politique de réhabilitation et d'amélioration de l'habitat. La politique de renouvellement urbain, quant à elle, est élaborée conjointement avec la ministre de la transition écologique, pour tenir compte des impératifs environnementaux. environnementaux. Le comité interministériel des villes qui s'est tenu au mois de janvier dernier a permis de mobiliser 3,3 milliards d'euros supplémentaires au bénéfice des quartiers prioritaires, dont plus de 1 milliard d'euros au titre du plan de relance. il a été décidé une hausse de 2 milliards d'euros des moyens dont dispose l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, portant ainsi son budget à 12 milliards d'euros pour le nouveau programme national de rénovation urbaine. Au travers de toutes ces politiques, l'État est présent pour garantir la cohésion des territoires, loin de l'image que certains se plaisent à véhiculer d'une France qui serait déchirée entre la ville, la banlieue et la campagne, d'une « France archipel », éclatée dans des espaces concurrents. Il nous faut aussi lutter contre cette vision erronée d'un État qui privilégierait les grandes métropoles, seules bénéficiaires des fruits de la croissance, au détriment d'une France périphérique qui serait oubliée- rien n'est plus faux ! Récemment, l'économiste Laurent Davezies a publié un ouvrage qui démontre que les inégalités territoriales n'ont pas explosé et que, sans l'État, certains territoires se seraient vidés. Il a montré, chiffres à l'appui, que l'emploi public a continué de progresser dans les départements dans lesquels l'emploi privé a reculé. Mais la présence des pouvoirs publics n'a pas toujours suffi à compenser des évolutions économiques profondes, comme la désindustrialisation. L'aménagement du territoire doit reposer aussi sur une économie prospère. Cela excède sans doute les termes du débat de ce jour, mais je tiens à le rappeler : avant la crise du covid-19, nous avions recommencé à créer de l'emploi industriel dans notre pays. Le plan France Relance nous permettra, dès cette année, de retrouver le chemin de la croissance, car il bénéficie en grande partie aux territoires. Ses crédits sont très largement territorialisés et seront déployés au travers des contrats de relance et de transition écologique. Le Premier ministre a souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner un projet de relance sur les domaines correspondant à ses besoins et ses objectifs. voilà ce que je tenais à dire en prélude à ce débat. En tant qu'ancien élu local- j'ai été maire d'une commune rurale et de montagne durant près de trente ans -, je sais qu'une politique d'aménagement du territoire ne peut se concevoir sans un dialogue constant avec les acteurs de terrain. C'est la raison pour laquelle le débat que nous allons avoir est non seulement utile, mais indispensable.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

À cet égard, les bureaux de poste jouent un rôle essentiel pour créer le lien entre La Poste, les habitants et les services dispensés. Force est de constater que La Poste est actuellement confrontée à une baisse de volume du courrier, estimée à 19 % pour l'année 2020. En effet, le service universel postal est devenu brutalement déficitaire de 1,5 milliard d'euros, alors qu'il était positif

tout de même rapporté à La Poste 300 millions d'euros cette année, ni par l'augmentation du prix du timbre. Faute de compensation financière par l'État, les missions de service public de La Poste risquent d'être mises à mal. Sont ainsi concernés non seulement le service universel postal, qui oblige La Poste à distribuer le courrier six jours sur sept, sur l'ensemble de notre territoire, mais également l'obligation de maintenir au moins 17 000 points de contact partout en France, malgré la fréquentation en baisse de 20 % des bureaux de poste en 2020. Dans cette perspective, La Poste entreprend sa modernisation : elle favorise la digitalisation, tisse des partenariats et assure la restructuration des bureaux de poste en fonction des besoins locaux. les bureaux de poste sont bien différents en fonction des territoires, ce qui provoque de nombreuses inquiétudes, notamment dans nos territoires ruraux. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre pour accompagner La Poste, afin de retrouver un équilibre budgétaire sans porter atteinte au maillage territorial ? Il est absolument nécessaire de garantir une présence sur l'ensemble de nos territoires, en particulier dans les territoires ruraux.

du tout le même poids dans le débat. Le service universel postal accuse un déficit massif depuis trois ans, porté à 1,5 milliard d'euros en 2020. Quant à la mission d'aménagement du territoire, qui se traduit par le maintien de 17 000 points de contact, elle n'est pas intégralement compensée. Mais le reste à charge pour l'entreprise n'est pas du même ordre

D'autre part, je suis comme vous très attaché au principe d'une implantation territoriale large de La Poste ; il ne faut pas que le réseau territorial subisse les contrecoups de la crise. Il est toutefois sain et nécessaire de s'assurer que le contrat de présence postale est toujours réaliste, en lien avec l'AMF, qui, avec l'État, en est signataire. En tout état de cause,

M. Ronan Dantec. Monsieur le secrétaire d'État, une étude publiée le mois dernier par l'Association des maires ruraux de France montre que les écarts en matière d'accès aux médecins généralistes ou spécialistes s'aggravent au détriment du monde rural. entières enregistrent des baisses spectaculaires de leur densité globale en médecins généralistes. S'ensuit une concentration des médecins restants sur les principaux centres urbains. Cette situation a des conséquences graves, qui peuvent se résumer en un seul chiffre : une

participent de cette évolution, qui s'aggrave chaque année. Il n'y a donc plus d'« égalité », pour reprendre votre terme, monsieur le secrétaire d'État, face aux soins dans notre pays. C'est un phénomène gravissime car, derrière, c'est aussi des entreprises qui ne s'installent pas et des familles qui préfèrent quitter un territoire où l'offre de soins est défaillante. Les déserts médicaux participent grandement du « désaménagement » du territoire exacerbent toutes les fractures territoriales et nourrissent la rancoeur qui s'installe chez nos concitoyens face à ce qu'ils considèrent être une démission du politique. La situation continue de se dégrader : des zones pourtant proches de grandes villes,

En écho aux propositions des réseaux de collectivités, envisagez-vous de vraies mesures non seulement incitatives, mais réellement contraignantes sur les installations, pour répondre enfin à ce qu'il convient d'appeler un scandale français

et d'instances de gouvernance de ces espaces, qui fédèrent, de part et d'autre de la frontière, nombre de niveaux de collectivités et d'institutions. Cela vise à faciliter, notamment sur ces territoires, la coordination des politiques d'aménagement. Les groupements européens de coopération territoriale en constituent la forme la plus aboutie,

Cependant, en pratique, de nombreux obstacles de nature juridique, administrative, linguistique, ainsi que des freins à la mobilité liés à des disparités économiques et aux différences socioculturelles continuent d'entraver la coopération transfrontalière. À cet égard, la mise à l'agenda politique du projet de loi 4D constitue une bonne nouvelle pour les territoires frontaliers ; l'idée de renforcer la décentralisation et la déconcentration leur offre des perspectives intéressantes, dans la mesure où ils côtoient des pays qui se caractérisent par un degré plus élevé de décentralisation et de déconcentration. Les acteurs de la coopération transfrontalière s'accordent pour dire que le projet de loi 4D s'inscrit dans la droite ligne de différentes initiatives qui doivent permettre de donner plus de marges de manoeuvre aux territoires, en particulier frontaliers.

? Quelles seront les mesures qui faciliteront la coordination des compétences de chaque niveau institutionnel au sein de nos espaces transfrontaliers, autour d'un même projet de développement territorial ? La

de la gestion des soins. La crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 a bien démontré l'intérêt d'une bonne coordination entre les autorités sanitaires françaises et celles des pays frontaliers. Il s'agit d'un enjeu majeur pour faciliter la vie des habitants et mieux organiser la coordination des soins sur un même bassin de vie,

Deuxièmement, pour renforcer la coopération en matière d'aménagement du territoire, nous proposerons probablement que les collectivités territoriales étrangères frontalières et limitrophes puissent être associées à l'élaboration d'un certain nombre d'éléments, dont les documents d'urbanisme. Actuellement, le code général des collectivités territoriales prévoit seulement des consultations au niveau régional ; il est possible d'en compléter les dispositions pour assurer la consultation de l'ensemble des autorités concernées par toutes les dimensions transfrontalières d'un bassin de vie. Troisièmement, nous envisageons d'autoriser les collectivités étrangères à participer au capital de certaines sociétés publiques locales, dès lors que leur objet social est exclusivement

un article publié le 11 juin 1982- son titre était : « Lozère : les enfermés du Gévaudan » -, évoquait la « pauvre nationale 88 ». On ne peut que regretter que sa modernisation ait si peu avancé depuis En 2018, Élisabeth Borne, alors ministre des transports, annonçait un effort inédit en matière d'infrastructures afin de contribuer à la cohésion des territoires. Lors de la présentation en conseil des ministres du projet de loi d'orientation des mobilités (LOM), un plan de désenclavement avait été évoqué : il portait sur une vingtaine d'itinéraires routiers jugés prioritaires, car structurants

dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à 2x2 voies ». La Lozère devrait donc bénéficier de cet effort. Le protocole de préfiguration du CPER 2021-2027 pour l'Occitanie, signé en présence de M. le Premier ministre à Tarbes, devrait en toute logique concrétiser cet engagement de l'État. Or il accorde peu de place à des investissements nouveaux sur les routes nationales. Cela vaut aussi bien pour la mise en 2x2 voies de la RN88 en Lozère que pour le contournement de Langogne, qui n'est toujours pas annoncé. Ma collègue Maryse Carrère pourrait vous dire exactement la même chose concernant la RN 21 entre Tarbes et Lourdes. Monsieur le secrétaire d'État, comment le Gouvernement envisage-t-il le financement des travaux d'aménagement de l'ensemble des routes nationales dont la RN88 ? Les protocoles de préfiguration vont-ils évoluer pour permettre le financement de ces travaux dans le cadre des le secrétaire d'État. Madame la sénatrice Pantel, vous m'interrogez sur la prise en compte des réseaux routiers dans le cadre des contrats de plan État-région en cours de négociation, singulièrement sur la situation de votre département et sur la nationale 88, laquelle a été

étape, marquant l'engagement coordonné de l'État et de la région. Il n'est pas un point final. En 2021, une large concertation avec les territoires permettra de préciser le contenu du

et tenir compte des démarches spécifiques en cours entre l'État et certains conseils régionaux, tels les protocoles sur des lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas. Monsieur le

être l'occasion de mettre en place une concertation accrue avec les élus de proximité, l'État poursuit sa démarche consistant à fermer les services publics : trésoreries, postes, gares, classes, voire écoles. Ces mesures successives ont mis en danger notre France rurale dans laquelle se battent nos agriculteurs, confrontés à la baisse insupportable de leurs revenus, tandis que les PME de proximité tentent de résister. Les collectivités territoriales, dont les finances et l'autonomie fiscale ont été malmenées, ont pour leur part du mal à répondre comme elles le souhaiteraient aux reste au coeur de nos préoccupations. Le département de la Dordogne compte 8,3 médecins pour 10 000 habitants, soit une densité inférieure à la moyenne régionale et nationale. Ces médecins, il faut le savoir, sont pour la plupart en milieu ou en fin de carrière, 35 % d'entre eux étant âgés de 60 ans ou plus. Cette désertification médicale a fortement réduit l'attractivité des territoires ruraux. Face à ce constat, la levée du n'aura pas d'effet à court terme,

Monsieur le secrétaire d'État, comment comptez-vous répondre à cette exigence d'égalité territoriale et redonner confiance à nos élus locaux, acteurs de proximité en première ligne en cette période de crise ? Que comptez-vous faire pour développer le réseau des centres de santé, qui permettent de mettre en oeuvre le droit à la santé de l'ensemble de nos concitoyens ?

Du fait de la crise sanitaire, de nombreux citadins envisagent de s'y installer. La loi dite 4D, c'est un fait, devra impérativement participer à la réduction des inégalités territoriales et sociales et nous y veillerons, monsieur le secrétaire d'État, car c'est une exigence, garante de la cohésion territoriale.

Je profite de cette occasion pour vous indiquer que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, que j'ai l'honneur de présider, organise un cycle d'auditions sur les perspectives de la politique de l'aménagement du territoire et qu'elle entend faire des propositions concrètes à moyen terme sur cette thématique. On pourrait aisément penser que ce débat est ancien, tout comme les nombreuses propositions déjà formulées par notre institution, mais il n'en est rien. D'une part, nous devons tous collectivement continuer à porter des propositions concrètes, reflétant notre expérience des territoires et de l'évolution de la politique d'aménagement du territoire

étant, je m'inquiète du manque d'effets visibles de ces politiques pour nos concitoyens. Comment comptez-vous assurer l'équilibre de notre territoire face à la puissance du phénomène de métropolisation, afin de permettre à chaque territoire de valoriser ses atouts ? Sur quel nouveau programme de cohésion travaillez-vous actuellement ?

de rapprocher l'offre de soins des besoins des populations. Quelles leçons tirez-vous des effets de la crise sanitaire actuelle sur l'organisation territoriale de notre système de soins ? La parole est à M. le secrétaire

programmes d'appui fonctionnent. Nous travaillons d'ailleurs à l'élaboration d'un nouveau programme, dont l'objet sera d'étendre les prestations d'ingénierie de l'ANCT aux communes de montagne. Il s'agira du premier programme de montagne depuis le plan Neige des années 1960-1970.

: « Dans cette période transitoire jusqu'à 2024, l'État travaille en étroite collaboration avec les collectivités chargées de la Gemapi, que ce soit pour les modalités de gestion de ces ouvrages, la réalisation de travaux de renforcement ou encore la préparation des dossiers d'autorisation de systèmes d'endiguement. Ces travaux ne seront donc plus à mener par les collectivités par la suite. » Or que constate-t-on réellement sur le terrain ? Des travaux insuffisants, un financement largement défaillant de la part de l'État et des collectivités dupées au regard de l'ampleur des coûts d'entretien.

vous alertaient déjà sur l'état des digues transférées. Monsieur le secrétaire d'État, êtes-vous aujourd'hui en mesure de rassurer les élus locaux sur la capacité de l'État à honorer ses engagements en matière de soutien financier ? Un fonds de compensation peut-il être envisagé pour mettre fin à l'inégalité de traitement entre digues domaniales et digues non domaniales, afin de consolider le système d'endiguement sur l'ensemble des bassins, et notamment celui de la Loire secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Bigot, vous m'interrogez sur la problématique spécifique de l'entretien des digues domaniales et sur les transferts de compétences aux collectivités à partir de 2024.

c'est-à-dire l'entretien, la surveillance, l'ingénierie et les travaux. Depuis le 1 janvier 2018, les EPCI sont devenus gestionnaires des ouvrages de protection. Afin de préparer la transition entre les anciens et les nouveaux gestionnaires, des périodes transitoires ont été prévues, notamment pour faciliter la mise en place des systèmes d'endiguement. C'est le cas notamment pour les digues de l'État.

pour la défense contre les inondations. Lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la loi Maptam, l'État, ou l'un de ses établissements publics, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'EPCI pendant une durée de dix ans, soit du 10 janvier 2014 au 28 janvier 2024.

Depuis plus de dix ans, une longue succession de renoncements, de demi-mesures de recentralisation, affirmées ou rampantes, se sont succédé, qui s'expliquent non seulement par les crises économiques successives ou par la métropolisation croissante, mais surtout par une réalité oubliée, que la crise sanitaire que nous traversons depuis un an est venue faire exploser.

Ce que la crise est venue nous rappeler, c'est que la question qui se pose est non plus celle des territoires, mais celle des gens. Il y a des gens, des personnes, des individus qui sont en droit de disposer d'un cadre de vie, d'un niveau de services, d'infrastructures leur permettant de vivre librement et en sécurité, bien souvent dans une belle fraternité d'ailleurs.

en matière hospitalière. Hors hôpital, la situation, vous le savez, n'est guère plus satisfaisante. Je rappelle que l'écart de densité médicale selon les départements varie de un à trois pour les généralistes et de un à huit pour les spécialistes. Je rappelle également que, aujourd'hui, entre 6 et 8 millions de Français vivent dans des déserts médicaux et que ce nombre n'a fait qu'augmenter au cours des dernières années. Cette situation a bien sûr des conséquences sanitaires, la carte des déserts médicaux se superposant à la carte de la mortalité précoce. À ce scandale sanitaire s'ajoute un scandale financier. Certaines estimations, notamment de la Cour des comptes, montrent que les dysfonctionnements en matière d'accès aux soins coûtent entre 1 et 5 milliards d'euros par an au contribuable.

Je m'inquiète toujours de son sort. Le Cerema accompagne les collectivités dans des démarches de coproduction permettant d'intégrer les enjeux nécessaires à la conduite du changement et d'apporter des réponses spécifiques adaptées aux contextes locaux. Or son plan de restructuration,

projets de loi 4D, Climat et résilience, ainsi que de l'adaptation au changement climatique, il n'est question pour le Cerema que de faire face à des baisses successives de moyens. Je m'interroge donc sur la volonté du Gouvernement de respecter les objectifs ambitieux du plan Biodiversité, initié en 2018, ainsi que la promesse d'un plan de relance orienté orienté vers la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, d'où ma question : comment mettre en pratique des politiques d'aménagement du territoire pour faire face au changement climatique en dégradant l'outil compétent et performant qui le permet ? monsieur le ministre, Cet organisme s'est doté d'un projet d'établissement permettant de recentrer son activité sur six domaines, tous liés à l'aménagement du territoire : mobilités ; infrastructures de transport ; environnement et risques naturels ; mer et littoral ; bâtiment ; ingénierie territoriale. L'adaptation des territoires au changement climatique est désormais le fil rouge de l'activité du Cerema. Centré sur des missions d'expertise en amont des projets de recherche et d'innovation, ainsi que de diffusion des connaissances, il agit en complémentarité avec l'ingénierie locale privée et publique, en particulier les agences techniques départementales. En tant que partenaire de l'ANCT, le Cerema intervient pour le compte de l'État et de 400 collectivités chaque collectivités chaque année, dont 80 collectivités de moins de 20 000 habitants. Il est porteur de sujets essentiels, tels que le programme national « France vue sur mer -Le sentier du littoral ». Il est aux côtés des territoires face à toutes les catastrophes, par exemple dans les vallées de la Roya et de la Vésubie à la suite de la tempête Alex. Il est là pour la sécurisation, la reconstruction transitoire

écologique (CRTE), qui ont naturellement une dimension rurale. Enfin, son système économique, fondé essentiellement sur une subvention pour charges de service public, lui permet d'intervenir en faveur de collectivités sur la base des modèles, grâce auxquels ces dernières bénéficient de quelques jours d'expertise gratuite, puis ne paient que 50 % environ du coût de la prestation si celle-ci

idée architecturale ne prend sens que s'il reste des maçons pour la concrétiser

En effet, l'activité économique est vitale pour les bassins de vie. C'est l'économie qui sous-tend le marché de l'emploi, le développement des services et la croissance démographique. Partout en France, nous avons des entreprises dans des secteurs de pointe qui marchent bien. Lorsqu'elles sont implantées en milieu rural, elles constituent des fleurons et, bien souvent, les principaux employeurs C'est par exemple le cas- je m'en excuse auprès de mes collègues, qui m'entendent de nouveau sur le sujet -, en Aveyron, de l'usine Bosch d'Onet-le-Château et de l'usine SAM de Viviez, au coeur de la Mecanic Vallée. Ces entreprises ont bénéficié d'aides publiques censées favoriser leur installation ou leur développement. On pourrait donc croire que l'aménagement du territoire fonctionne bien. Pourtant, les annonces de presque 1 000 suppressions d'emplois et l'arrêt des chaînes de production sur les deux sites aveyronnais voilà deux semaines

Voilà trois mois encore, j'alertais le ministre de l'économie sur les conséquences des mesures prises au nom de la transition écologique pour les filières industrielles. Alors que, en 2019, le ministre se déclarait favorable à ce que les nouveaux véhicules diesel moins polluants puissent être éligibles à la vignette Crit'Air 1, il a exclu en janvier 2021 les véhicules hybrides diesel des aides à l'achat des voitures neuves. neuves. Résultat, en Aveyron, trois mois plus tard, nous pouvons constater les conséquences du choix idéologique de la désindustrialisation concernant la filière automobile diesel en France. Cet échec, c'est aussi celui de l'aménagement du territoire à la française. L'exemple montre bien les effets ravageurs et en cascade de telles décisions politiques. Elles nécessitent plus de prospective. Monsieur le secrétaire d'État, comment le Gouvernement envisage-t-il de réindustrialiser la France ? Comment faire pour que la réindustrialisation du territoire se conjugue durablement avec son aménagement ?

territoires d'industrie recouvrant près de 500 intercommunalités ont fait émerger 1 500 projets d'investissements concrets, dont 57 sont déjà déployés. Le programme a été renforcé dans le cadre du plan France Relance,

Si j'avais pu avoir un temps d'échanges avec vous, je vous aurais volontiers dit deux ou trois choses de ce territoire particulier, notamment que nous manquons de médecins, surtout de spécialistes. Aménager le territoire, c'est garantir l'égalité d'accès aux soins, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que toute Française puisse avoir accès à un gynécologue. Or, sur ce territoire de 48 000 habitants, il n'y en a qu'un seul ! La moyenne française étant de 17,6 pour 100 000 habitants, il nous en faudrait

Il en résulte notamment de graves manques dans le suivi de santé des femmes. Les déserts médicaux ne sont pas une vue de l'esprit ; ils sont une triste réalité. L'Occitanie, région pourtant attractive, est passée en dix ans d'une situation de surdotation à une situation de sous-dotation en professionnels de santé. Alors que nous manquons de praticiens et que le nombre de seniors dépendants devrait augmenter de 60 % en cinq ans, 70 % de ces médecins partiront à la retraite d'ici à 2026. Or les jeunes médecins, et leur choix parfaitement respectable, n'assurent pas toujours le même nombre de consultations. Si l'on ne remplace que les départs à la retraite, la fracture sanitaire va continuer à s'accentuer. La formation des médecins est dispensée par les établissements publics d'enseignement supérieur et est quasiment gratuite. Le coût moyen de formation d'un étudiant en médecine est d'environ 150 000 euros. Pourtant, les praticiens continuent de s'installer dans des zones surdotées quand l'État et les collectivités territoriales investissent dans les territoires sous-dotés. L'aménagement du territoire n'implique-t-il pas de répondre aux besoins des habitants, dont la santé n'est pas le moindre, et de faire en sorte de les satisfaire ? Où en est-on, par exemple, du déconventionnement ? La parole

Alors que le projet de loi Climat et résilience va faire son entrée dans l'hémicycle de la Haute Assemblée, de même bientôt- nous l'espérons -que le projet de loi 4D, il est important de penser à l'avenir de nos espaces ruraux. Si lutter contre l'artificialisation des terres est une nécessité partagée pour préserver ce bien commun qu'est notre environnement, il n'en demeure pas moins que nos espaces ne doivent pas être mis sous cloche et qu'il nous faut chercher un juste équilibre entre protection et dynamique de nos territoires ruraux. Or les outils mis en place jusqu'à présent par les politiques de l'État ne répondent qu'à un seul objectif : réduire, voire interdire l'utilisation de l'espace. Comment concevoir dès lors une ruralité attractive, vivante, dans la mesure où aucune solution autre que l'interdiction de construire n'est vraiment proposée ? La crise sanitaire a confirmé l'engouement des Français à voir dans les campagnes l'accès à une meilleure qualité de vie. Alors que les villes manquent cruellement de logements, il existe un fort potentiel, sans construction nouvelle, dans les communes rurales, dont certaines souffrent de désertification. N'y aurait-il pas ici une occasion à saisir ? Dans mon département, les Alpes-Maritimes, la petite commune d'Ascros a sauvé son école en lançant un appel pour que de nouvelles familles viennent s'installer dans des logements vacants de son village. Cela a été du gagnant-gagnant. Mais une telle initiative est malheureusement trop rare. Monsieur le secrétaire d'État, un grand nombre de maires ruraux comptent sur la mise en oeuvre d'un plan national ambitieux de résorption de la vacance et de transformation ou de rénovation de bâtis inoccupés pour revitaliser nos campagnes et accueillir des actifs. Qu'en pensez-vous ?

intercommunalité soient couvertes par des opérations de revitalisation de territoire (ORT). Celles-ci permettent en particulier de mettre en place l'avantage fiscal dit « Denormandie ancien » pour les Français qui souhaitent investir dans nos territoires en rénovant des logements, de renforcer le droit de préemption urbain et de faciliter l'installation et la rénovation des commerces. C'est évidemment intimement lié à l'attractivité des logements, donc à l'envie des Français de s'installer dans ces territoires. Les ORT peuvent bénéficier à

des projets d'aménagement. Nous avons également mobilisé d'importants moyens financiers dans le plan de relance, qui prévoit 300 millions d'euros pour combler les déficits des opérations de recyclage ou de rénovation d'îlots bloquant fortement les opérations. Les remontées en cours sont importantes. Le plan connaît d'ailleurs un franc succès. Je mentionne également le plan de lutte contre la vacance, qui concerne tous les territoires et qui vise à outiller les collectivités pour recenser les logements vacants et les outils disponibles aux échelons national et local et accompagner ainsi les propriétaires.

aux maires. Ces derniers sont dépourvus face à ce véritable fléau qu'est la vacance de logements en milieu rural. La

l'annonce d'un véritable renouveau de cette coopération, qui semblait en panne de volonté politique du côté de la France. Pourtant, deux cadres existent, et ils pourraient être mieux exploités.

Ce groupement européen de coopération territoriale rassemble une zone plus resserrée : le département des Pyrénées-Orientales et la province de Gérone. Beaucoup a déjà été fait pour permettre aux habitants de profiter d'équipements en commun. Je pense notamment à l'hôpital franco-espagnol de Cerdagne, exemple unique en Europe, à la station d'épuration des eaux usées sur le Sègre, affluent de l'Èbre, ou à l'abattoir transfrontalier d'Ur ; le domaine culturel n'est pas en reste, puisque nous avons plusieurs parcours transfrontaliers de routes patrimoniales. tant reste à faire ! Monsieur le secrétaire d'État, la loi 4D inclura-t-elle des dispositions facilitant les coopérations entre les cantons et les villes de part et d'autre de la frontière, afin de permettre aux habitants d'accéder à plus d'équipements communs, comme une université transfrontalière ? monsieur le ministre,

le sujet. Je vous remercie d'avoir souligné la volonté politique affichée lors du sommet du 15 mars dernier en faveur du renouveau de la coopération transfrontalière franco-espagnole. Nous sommes plus qu'attentifs au développement des territoires qui bordent la frontière espagnole sur

Il y en a beaucoup d'autres à l'échelle locale ; nombre d'entre elles s'inscrivent dans le cadre de programmes européens. D'ailleurs, je remercie vivement les élus de leur implication dans ces structures de coopération transfrontalière. La déclaration du 15 mars appelle une amplification de la dynamique et prévoit le lancement d'un travail conjoint pour une nouvelle stratégie franco-espagnole sur cette frontière. Les sujets ne manquent pas. Bien entendu, il s'agit des passages transfrontaliers, qu'il faut décongestionner par de nouvelles solutions ne passant pas seulement par les deux extrémités des frontières. Ainsi, la mutualisation d'équipements peut être développée en surmontant quelques obstacles juridiques et administratifs. Vous avez

nous avons la chance d'avoir un secrétaire d'État chargé de la ruralité, je crois que vous feriez oeuvre utile en faisant en sorte que même les ruraux, dans l'attente de la 4G et de la 5G, puissent accéder au télétravail et, tout simplement, au service universel ! La parole

Les villes sont de plus en plus bétonnées, embouteillées, tandis que les territoires ruraux sont de plus en plus isolés et abandonnés. On ferme des classes, des services postaux, des guichets ... Personne ne s'y retrouve. Face à cela, soit on continue avec le « tout-métropole », soit on fait en sorte que nos villes redeviennent des locomotives, et non des aspirateurs ! Pour cela, il faut créer des emplois, faire venir des habitants et s'appuyer sur une démarche raisonnée de développement de nos transports en commun et de nos infrastructures numériques. Je pense évidemment en particulier à la fibre optique. Il ne s'agit pas, bien sûr, de plaider pour « la petite maison dans la prairie » ou l'étalement urbain, mais d'accompagner une démarche raisonnée de développement de nos villes moyennes et de nos centres-bourgs. Monsieur le secrétaire d'État, êtes-vous prêt à prendre ce tournant ? Les Français vous le demandent, ils aspirent à des communautés plus réduites, plus humaines, à plus petite échelle ; notre société est fragile, la violence augmente partout, l'aménagement du territoire est un vrai levier pour lui redonner un peu de cohésion. La parole

Un rapport récent de l'Institut Montaigne indique que les quinze métropoles de plus de 500 000 habitants représentent plus de 50 % de l'activité économique et qu'elles captent les secteurs les plus porteurs de croissance. C'est indéniable. L'action des pouvoirs publics doit en tenir compte pour assurer la cohésion des territoires, mais aussi le bien-être des habitants qui subissent l'augmentation du prix de l'immobilier dans des secteurs concentrant, en plus, des emplois. Ce sujet n'est d'ailleurs pas perçu partout de la même façon dans les territoires. Je me suis rendu il y a très peu de temps dans les monts du Lyonnais pour labelliser des « petites villes de

De toute évidence, et nous en prenons acte, le contexte connaît des transformations profondes : mondialisation économique accentuant la métropolisation, décentralisation, construction européenne. De nouveaux sujets apparaissent, comme le développement durable ou le numérique, qui modifient le sens et le contenu de cette politique. Le constat est simple, Didier Mandelli l'a souligné, la photographie de la France métropolitaine en 2021 est celle d'un pays où quinze métropoles polarisent le développement économique pendant que les « territoires épars », qui représentent 90 % de la superficie et 70 % de la population du pays, voient leur croissance et leur niveau de vie stagner, voire décliner. Nous avons bien conscience que le développement de pôles d'attractivité économique, démographique, culturelle de dimensions européenne et mondiale, constitue un atout indéniable pour la France. Pour autant, un tel développement, au détriment de certains territoires toujours plus marginalisés, doit être interrogé. Seule une politique volontariste permettra de réussir ce rééquilibrage. Elle devra s'inscrire dans la perspective d'un renforcement durable et structurel de l'attractivité économique des territoires ruraux. Dès lors, il est nécessaire de repenser l'action publique en favorisant la différenciation selon les territoires et, ainsi, de renforcer durablement la cohésion à l'échelle nationale, dont l'État est garant, en mobilisant toutes les parties prenantes. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons en a été un puissant révélateur. C'est désormais selon cet axiome que doivent être pensées les différentes actions de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Ces actions conféreront à ces dernières une confiance renforcée,

mise en avant au sein de l'agenda rural ; elle doit être systématiquement préférée, car elle offre de la cohérence grâce à la prise en compte de la décentralisation et des spécificités locales. C'est la condition d'un aménagement du territoire concerté et mobilisateur pour tous. Il nous faut retrouver aussi la raison d'être de l'aménagement du territoire : obtenir un véritable effet contracyclique par rapport aux déséquilibres spontanément créés par les forces de concentration autour des grandes aires urbaines, et pondérer les disparités en termes d'isolement ou de revenu par habitant. Pour y parvenir, il faut réellement organiser la métropolisation afin que celle-ci bénéficie au plus grand nombre. L'objectif de rayonnement reste cependant peu concret, ainsi que le souligne le tout récent rapport de la Cour des comptes pour 2020. D'autre part, il faut soutenir plus intensément les réels leviers d'émancipation et d'attractivité des territoires que sont le développement d'une offre de formation universitaire et professionnelle couverture numérique pérenne et homogène accompagnée d'une réelle pédagogie, et relever le défi de l'écomobilité. Enfin, il faut véritablement s'atteler à une action renforcée de l'ANCT- c'était l'une des propositions de notre

L'Agence, en fluidifiant et en rationalisant l'existant, doit permettre aux territoires moins denses de se développer grâce à des projets propres, sans voir leurs potentialités aspirées par d'autres territoires plus aguerris. En conclusion, je ne peux que réitérer avec force ce que nous disions déjà dans notre rapport et qui reste particulièrement d'actualité : il faut rétablir un État stratège, régulateur, véritable pilote de la politique d'aménagement du territoire autour des binômes région-intercommunalité- acteur majeur -et département-commune. Le critère d'aménagement du territoire doit être prioritaire dans les choix de régulation et d'investissement de l'État, lequel doit cesser de fonctionner en silos et envisager sa politique comme un projet global et prospectif. La crise actuelle ne nous laisse plus le choix. Favoriser les territoires les plus compétitifs pour attirer les entreprises et créer de l'emploi, d'une part, et maintenir une offre de service public dans tous les territoires et pour tous les habitants, d'autre part, ne sont pas nécessairement deux approches contradictoires.

un grand port de commerce. Et puisque nous sommes ici au Palais du Luxembourg, n'oublions pas que c'est sous Louis XIII que fut constituée la marine d'État.

Tout allait donc bien, et les activités se sont développées jusqu'à la décision des Britanniques, en 2016, de quitter l'Union européenne.

maritime est particulière car, au transport maritime, très ancien, s'est ajouté depuis 1994 le ferroviaire, avec le tunnel sous la Manche. Le Gouvernement partage bien évidemment vos préoccupations quant à l'avenir des liaisons entre la France et le Royaume-Uni.

Le constat est clair : si le secteur du transport global- maritime, terrestre, aérien ; je n'oublie pas ce dernier segment -a été touché par la crise de manière hétérogène, le transport sur et sous la Manche a, quant à lui, été très fortement impacté. Les transports opérés sous pavillon français par Brittany Ferries et DFDS Seaways ont connu au printemps 2020 des baisses de fréquentation de passagers jusqu'à 80 % et des pertes de chiffre d'affaires de 75 % par rapport à 2019. Il en est de même pour le tunnel, plus spécifiquement pour l'Eurostar, qui a connu des baisses dans des proportions identiques. Les mesures sanitaires prises de part et d'autre de la Manche depuis un an empêchent pour le moment la reprise du trafic, mais le gouvernement français n'est pas inactif. L'État a toujours été aux côtés des opérateurs durant la crise et il le demeurera le temps qu'il faudra, au principe du « quoi qu'il en coûte ». Souvenons-nous des paroles du Président de la République, qui concernent évidemment les transports. Les dispositifs d'aide d'urgence,

avec les organisations syndicales, diminuer le temps de travail et pratiquer la modération salariale, à condition de maintenir intégralement l'emploi. L'État a porté, dès le début de la crise, une attention toute particulière aux compagnies de ferries, touchées de plein fouet par les mesures de confinement et de restrictions des déplacements.

Les infrastructures nécessaires au rétablissement des contrôles aux frontières ont été installées. Tous les ports français des Hauts-de-France, de Normandie ou de Bretagne ont su anticiper la date de sortie

Face au lancement, en novembre dernier, par le gouvernement britannique d'une procédure d'appel d'offres pour la création de dix ports francs, la France ne va pas rester sans réponse. Le Président de la République a souhaité que nous nous engagions. Une réflexion a été entreprise pour renforcer l'attractivité de nos zones industrialo-portuaires et une mission a été lancée afin d'étudier la mise en place de dispositifs permettant d'améliorer leur compétitivité. Le transport ferroviaire n'est pas en reste : Eurotunnel a investi 48 millions d'euros pour le rétablissement des contrôles frontaliers. Le Brexit crée aussi de nouvelles opportunités

S'agissant, enfin, du service Eurostar, le bouclage du plan de sauvetage passe avant tout par un effort des actionnaires et une plus grande implication des banques. Les discussions sont en cours. Le gouvernement français est prêt, s'il le faut, à prendre sa part, mais dans un effort partagé avec le Royaume-Uni. Enfin, je souhaite évoquer trois sujets majeurs. Je parlais d'opportunités à venir. J'ai lancé la semaine dernière la seconde phase du Fontenoy du Maritime. Depuis octobre, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs sur la compétitivité de notre marine marchande. Cet exercice doit aboutir, avant l'été,

mais en tant que ministre de la mer, je souhaite que notre pays soit une grande puissance maritime. Cela passe notamment par une véritable politique publique du, qui nous a longtemps fait défaut. Le Fontenoy du Maritime répondra à cette ambition. Je parlais d'une action déterminée de l'État :

de la manière la plus concrète aux attentes des acteurs économiques. Les acteurs du portuaire peuvent ainsi bénéficier de 200 millions d'euros pour accélérer la transition écologique et le report modal, deux dimensions clés

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé. Dans le débat

près d'un quart des émissions mondiales, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les transports ont une lourde responsabilité dans les bilans carbone nationaux et internationaux. Si la circulation maritime ne représente qu'une petite part de ce volume,

D'autres technologies apparaissent, comme la propulsion vélique, l'électrification des quais, le recours à des carburants alternatifs, le gaz naturel liquéfié (GNL) et, surtout, l'hydrogène. Pour financer ces nécessaires innovations, la création d'un fonds maritime vert comme mécanisme de suramortissement pour tout investissement vert dans la flotte ou encore l'instauration- enfin ! -d'une taxe carbone sur les carburants marins et aériens doivent être mises en débat. débat. Madame la ministre, ma question est multiple. Quelle transition énergétique est-elle prévue pour le transport maritime de voyageurs afin de réduire l'empreinte environnementale des bateaux ainsi que leur consommation ? Pour ce faire, quels projets peuvent être développés conjointement avec l'Angleterre, comme nous avons su le faire avec Eurotunnel ? Quel portage comptez-vous faire de cette question au niveau européen et, plus largement, à l'international, étant entendu que seules des actions globales peuvent avoir des impacts significatifs sur ces sujets ? Mme la ministre. Monsieur le sénateur Jacques Fernique, je connais votre intérêt pour cette problématique, puisque vous êtes membre de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. La transition énergétique du transport maritime va nécessiter des coopérations internationales,

mon ministère porte la charte Sails qui vise à limiter l'utilisation des carburants à fort taux de soufre, mais aussi à adapter la navigation dans les aires marines protégées et à sensibiliser les passagers au respect de l'environnement. Aujourd'hui, 14 compagnies ont déjà signé

Madame la ministre, le secteur maritime trans-Manche est doublement affecté, par le Brexit et par la crise du coronavirus. Il accuse sur l'année 2020 un recul de 80 % de son chiffre d'affaires. L'activité de transport de passagers à ce jour est quasiment inexistante et sans aucune perspective de reprise. Brittany Ferries est la compagnie la plus touchée par la crise : de 2,5 millions de passagers, elle est passée à 700 000 en 2020.

la compagnie a bénéficié d'un PGE à hauteur de 117 millions d'euros. En septembre 2020, notre Premier ministre a déclaré que le Gouvernement allait encore accentuer son soutien à la compagnie finistérienne en procédant au remboursement de ses charges sociales pour l'exercice 2021. Cet engagement porte sur un montant de 15 millions d'euros. Les acteurs économiques du trans-Manche ont acté le principe selon lequel la crise traversée allait structurellement bouleverser leur secteur d'activité.

-est un enjeu fondamental face aux avantages concurrentiels dont bénéficient certains pavillons par rapport au pavillon français. Une pérennisation du dispositif de remboursement des charges sociales tout au long de la durée de remboursement des PGE ou,, jusqu'à la fin de la crise sanitaire, pourrait à ce titre être débattue dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement la sécurité sociale pour 2022. Madame la ministre, ma question porte sur l'engagement pris par le Premier ministre de procéder au remboursement des charges sociales pour l'exercice 2021. Pouvez-vous nous indiquer la date de parution du décret permettant ce remboursement ? La parole

avec plus de 5 000 kilomètres de linéaire côtier métropolitain, la France peut s'enorgueillir de posséder l'une des plus grandes façades maritimes d'Europe. Pourtant, le trafic de nos principaux ports se place loin derrière celui de nos voisins. du Havre, premier port à conteneurs français, ne représente que le quart, voire le cinquième, de celle de ports comme Rotterdam, Anvers ou Hambourg. Si l'on considère les données en tonnage de marchandises, les résultats ne sont guère différents. différents. Avec ses 65 millions d'habitants, la France représente la part la plus importante du marché européen après l'Allemagne. Un avantage compétitif ne se bâtit pas en un jour. Cela nécessite des investissements massifs sur le long terme dans les infrastructures et la logistique. Certes, cette différence constatée peut aussi être en partie liée à la géographie. Toutefois, un tel déséquilibre interroge. Ma question est donc la suivante, madame la ministre : quelle est la stratégie du Gouvernement pour le développement économique de nos littoraux, en particulier de nos ports ? Alors que nous sommes à un tournant de la mondialisation du fait des évolutions socio-économiques, de la montée des préoccupations environnementales, de la crise sanitaire et du Brexit, vers quel secteur devons-nous concentrer nos efforts ? Il peut s'agir aussi bien du commerce de marchandises, des activités industrielles dans les zones portuaires ou de la politique de pêche que du transport de passagers et du développement touristique. Mon interrogation découle du sentiment général que notre pays ne tire pas suffisamment parti du potentiel que représente sa façade maritime exceptionnelle. Vous l'aurez compris, ma question ne se limite pas strictement à celle, tout à fait légitime, des liaisons trans-Manche. L'objectif est d'essayer de réfléchir également, à plus long terme, à la façon dont la mer peut s'inscrire dans notre trajectoire de redressement économique.

Brulin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire et le Brexit fragilisent terriblement le trafic trans-Manche. Pourtant, plus la situation se dégrade et moins vous semblez vous intéresser à la situation des liaisons maritimes. L'activité partielle et les prêts garantis ont certes été activés, mais aucune aide spécifique n'a été à ce stade

Les remboursements de cotisations sociales et salariales que vous avez évoqués ne sont pas encore effectifs, et il faudra manifestement attendre quelques mois encore pour qu'ils le soient. De plus, la ligne Dieppe-Newhaven, opérée par DFDS Seaways dans le cadre d'une délégation de service public (DSP), en serait exclue. Rien dans le plan de relance, rien non plus dans les contrats de plan État-région, notamment en faveur de nos ports. Quant au fonds de compensation du Brexit, la France ne touchera que 421 millions d'euros sur plus de 4 milliards au total. De plus, ce dernier ne prend en charge que les dépenses de l'État, à l'exclusion les collectivités. Tel est le premier sujet sur lequel je souhaite vous interpeller, madame la ministre. À cela s'ajoute que la filière devrait mettre en oeuvre dans moins d'un an de nouveaux dispositifs très complexes décidés par l'Europe pour ses frontières externes, afin de réaliser des contrôles biométriques avec le système

Envisagez-vous de plaider auprès de l'Union européenne un report de la mise en place de ce système ? Quel plan de promotion des traversées comptez-vous développer ? Telles sont quelques-unes de mes questions, madame la ministre. La concurrence étant très forte dans ce secteur, il est urgent d'apporter un soutien concret et réel au trans-Manche.

l'emploi maritime. Vous m'avez également interrogée sur l'EES, c'est-à-dire le système des entrées/sorties qui a été instauré par l'Europe

les entreprises du trans-Manche sont aujourd'hui victimes d'une situation exceptionnelle à double titre, du fait du Brexit et de la mise en place de mesures sanitaires strictes à la frontière du Royaume-Uni. Dans le Pas-de-Calais, les entreprises privées assurant la liaison trans-Manche emploient plus de 10 000 personnes, et bien davantage à l'échelon national. Aujourd'hui, ces entreprises

de la covid qui a conduit à fermer la frontière de la Grande-Bretagne plus que toutes les autres, comme pour sanctionner une nouvelle fois les Britanniques de leur départ de l'Union européenne, alors que finalement, c'est nous qui souffrons. Certaines entreprises ont déjà présenté leur plan de licenciements ; d'autres, comme Eurotunnel, cherchent à maintenir l'emploi en attendant une réponse gouvernementale à la hauteur des enjeux. De plus, dans la continuité de l'accord Brexit, il est impératif de contrôler l'effectivité du protocole nord-irlandais repoussé unilatéralement au mois d'octobre 2021, ce qui détourne la frontière et constitue une concurrence déloyale inacceptable à l'entrée du territoire européen. Il est très important que le Gouvernement établisse un dialogue constructif et direct avec le Royaume-Uni. Pour la suite, des propositions concrètes existent : un véritable plan de relance des entreprises du trans-Manche, et plus largement, des emplois logistiques et touristiques de la façade Manche-Mer du Nord la mise en place du pour le tunnel et les ports, qui ne dépend plus que de l'autorisation du Gouvernement car la Commission n'a pas émis d'objection ; la simplification des conditions de voyage vers la France pour les Britanniques vaccinés le redémarrage du trafic Eurostar par le soutien de l'État avec, en contrepartie, des arrêts à Calais-Fréthun, nouvelle porte d'entrée de l'Union européenne. Qu'attendons-nous encore pour mettre en place ces mesures de bon sens ? La

principalement en raison de la crise sanitaire. Son chiffre d'affaires a chuté en 2020 de 75 % par rapport à 2019. Malgré la mise en place d'un prêt bancaire de 450 millions d'euros en juin dernier et l'aide des actionnaires à hauteur de 210 millions d'euros, le maintien des restrictions de circulation fait craindre une nouvelle crise de liquidités dès le deuxième semestre 2021. Nous y veillons et nous y travaillons.

La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte. Madame la ministre, comme l'a indiqué Jean-Marc Roué, président du conseil de surveillance de Brittany Ferries, lors de l'assemblée générale de la semaine dernière, la crise sanitaire s'ajoutant à celle du Brexit a frappé la compagnie trans-Manche d'une double peine. Celle-ci lutte avec beaucoup de difficulté depuis un an pour préserver les emplois et maintenir son activité. Mais à l'heure où la contamination est loin d'être maîtrisée dans toute l'Europe, et même si la campagne de vaccination bat son plein et que les mesures sont drastiques,

est-il envisageable que la nouvelle stratégie vaccinale esquissée par le Président de la République, et ciblée sur des professions exposées, soit ouverte à d'autres secteurs les plus en contact avec la population, à l'exemple des salariés du trans-Manche ? La parole est à

Voilà presque trois mois que le Royaume-Uni est définitivement sorti de l'Union européenne. Les entreprises du trans-Manche, tout comme les ports de la façade Nord-Ouest, qu'ils soient situés dans les Hauts-de-France, en Normandie ou en Bretagne, n'ont pas attendu la date fatidique du 1 janvier dernier pour anticiper cette nouvelle réalité. acteurs ont montré leur capacité de résilience et d'adaptation aux conséquences de cette séparation. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est la crise sanitaire qui entraîne un choc supplémentaire et concomitant. Les acteurs du trans-Manche subissent ainsi la double peine- Brexit et covid-19 -, sans oublier la concurrence des grands ports du nord de l'Europe. Ils sont aujourd'hui très inquiets et dans une situation critique. Une réserve d'ajustement au Brexit est prévue pour en atténuer l'impact et soutenir les secteurs les plus touchés. Face à l'injuste répartition de cette réserve que propose la Commission européenne, j'ai appelé avec mon collègue Christian Cambon un rééquilibrage de cette enveloppe au profit de notre pays et, par conséquent, de l'ensemble des collectivités et entreprises concernées. Les opérateurs du trans-Manche- je tiens à insister sur le rôle et la place des ports dans ce système -doivent pouvoir bénéficier de ces fonds pour couvrir les dépenses d'aménagement requises par le retrait britannique. Je rappelle que 70 % des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne transitent par le Nord de France.

très en amont par les opérateurs seront couvertes par la réserve d'ajustement Mme la ministre. Monsieur le député Jean-François Rapin, vous avez raison de souligner que la France dans sa globalité, le Gouvernement, mais aussi les collectivités et l'ensemble des acteurs économiques ont anticipé

Aussi incroyable que ce soit, après plus de quatre années de négociations complexes, ces mots sont parfois prononcés dans les Hauts-de-France dès que l'on approche le port de Dunkerque et son écosystème. Le territoire dunkerquois a compris très tôt l'importance qu'allait revêtir le départ des Britanniques sur la relation trans-Manche et l'économie en résultant. J'ai eu de nombreux échanges avec les acteurs de terrain, particulièrement les autorités portuaires et les entreprises. a été très bien organisée. Je salue la capacité d'adaptation et la réactivité dont chacun a su faire preuve. Les services de l'État, notamment douaniers, ont mis en place un accompagnement efficace. Le port de Dunkerque a transformé son activité, réorganisé sa distribution et anticipé tous les cas de figure. L'annonce de l'accord de commerce et de coopération fut, tout de même, un soulagement pour nos entreprises. Le port a saisi les opportunités qui s'offraient à lui, et il devrait prendre prochainement la place de premier port européen pour le trafic avec l'Irlande.

L'Europe doit pouvoir se défendre et rester unie. À cet égard, la flexibilité importante des ports belges ou encore hollandais, tout comme la création de ports francs en Angleterre, ne peuvent que nous interpeller.

de la Seine-Maritime, sous forme d'une DSP, génère 48 millions d'euros par an de retombées à l'échelle départementale, 82 millions d'euros à l'échelle régionale et 219 millions d'euros à l'échelle nationale. Or il ne s'agit pas de la plus importante des lignes trans-Manche.

Les liaisons trans-Manche ne figurent pas dans le du Brexit, ce qui suscite une incertitude quant à leur avenir. Il n'est pas certain que les collectivités aient encore le droit d'aider financièrement les entreprises de ferries comme elles l'ont fait jusqu'à

Par ailleurs, un équilibre non coopératif se met en place. Les Anglais achètent aux compagnies des capacités de transport pour leurs approvisionnements vitaux, les faisant ainsi bénéficier d'une forme de soutien au détriment des besoins de transport français. Enfin, le Brexit peut être une occasion de rééquilibrer la situation. En effet, pour l'instant, les lignes profitent aux deux pays, mais ne sont soutenues financièrement que par la France. Dans ces conditions, madame la ministre, allez-vous négocier avec la Grande-Bretagne des accords spécifiques sur les liaisons maritimes trans-Manche ? La parole est à Mme

À ce stade, la France a choisi- je l'ai précisé lors de mes interventions précédentes -d'apporter un soutien économique direct aux armateurs, tant par le biais des mesures de droit commun que j'ai citées que par celui de dispositifs spécifiques. Ce choix de soutenir les compagnies

aujourd'hui que 2 % de l'activité. La baisse de volumes touche aussi le fret, après une légère embellie à la fin de 2020, alors que les Britanniques constituaient des stocks. Cette situation précipitera les compagnies sur les rochers, tout droit vers le naufrage, si des mesures fortes ne sont pas prises. Tous les opérateurs ne partagent pas nécessairement votre optimisme. DFDS Seaways a engagé un premier plan social qui prévoit le départ de 152 personnes sur les sites de Calais et Dieppe, par redéploiement et départs volontaires, avec heureusement un seul licenciement.

évoquer l'avenir des entreprises assurant les liaisons trans-Manche sans mentionner la situation de la compagnie Brittany Ferries. Créée en 1972 par des bâtisseurs visionnaires, soucieux de désenclaver leur territoire excentré, la compagnie finistérienne est devenue au fil des ans le premier transporteur maritime dans la Manche ouest et centrale, et le premier employeur de marins français. Les restrictions sanitaires liées à la pandémie de covid-19 ont très fortement réduit le trafic de passagers depuis un an, affectant ainsi la santé économique des opérateurs. Dès le 21 avril 2020, sur la proposition de Pascal Allizard, Philippe Bas et Jean Bizet, nous alertions le Premier ministre sur la nécessité de mettre en place un plan d'action volontariste et ambitieux pour une filière qui, avant la crise sanitaire, était déjà dans la crainte des effets du Brexit.

Dans un courrier de réponse, le 30 septembre dernier, M. le ministre délégué chargé des transports rappelait que le Gouvernement s'était engagé à attribuer aux compagnies une subvention correspondant à un remboursement de charges salariales

et des subventions de portage pour 20 millions d'euros. Telles sont les propositions que nous avons faites à la Commission européenne.

L'enjeu est en effet de taille puisque près de 6 millions de camions transitent chaque année entre les ports de la région des Hauts-de-France et la Grande-Bretagne, ce qui représente 70 % des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. le site de Calais voit ainsi passer 4 millions de camions les ferries et le tunnel, et son port reçoit environ 40 millions de tonnes de marchandises par an. L'entrée en vigueur du Brexit et la mise en place de nouvelles procédures et obligations douanières, vétérinaires et phytosanitaires ne sont pas sans conséquence sur la fluidité du trafic. Des ralentissements dus aux contrôles à la frontière ont été observés au début de l'année, malgré la création par les services de la douane française, en collaboration avec le port de Calais, les opérateurs maritimes et ferroviaires et les services de l'État, d'une frontière dite « intelligente » reposant sur l'utilisation des nouvelles technologies. Certes, des investissements ont été faits par les opérateurs trans-Manche et l'État à hauteur de 40 millions d'euros, dont 12 millions ont été apportés par le port Boulogne Calais

tenu des remontées de terrain et des constats effectués à la fois par les professionnels, les transporteurs et les services de l'État, quelles mesures comptez-vous prendre pour assurer la fluidité du lien trans-Manche et éviter l'engorgement de l'autoroute A16 ? En parallèle se pose la question du développement du ferroutage.

des flux entre le nord et le sud de l'Europe. La création d'une ligne de fret ferroviaire entre Sète et Calais a, quant à elle, été confirmée en juillet dernier, ce qui assurera une liaison notamment pour les containers maritimes. De quelle manière le Gouvernement compte-t-il accompagner ce type de projet permettant aux transporteurs de disposer de solutions de report modal au sein même du port ?

est surtout un lien maritime incontournable au coeur de l'entente cordiale entre nos deux pays, entente souvent tumultueuse que le Brexit a de nouveau fragilisée, notamment pour ce qui est des relations maritimes. L'annonce en novembre 2020 de la création de dix ports francs au Royaume-Uni a ravivé les tensions des deux côtés de la Manche. Le choix des huit premiers sites retenus, le 3 mars dernier, pour devenir les premiers ports francs géographiques d'Europe a donné corps à l'ambition anglaise. Madame la ministre,

élue de la Porte Océane, vous connaissez mon attachement à l'essor des grands ports maritimes. Le Havre doit naturellement jouer un rôle dans les relations trans-Manche et occuper une place prépondérante. Conscient de cette nécessité, l'État s'est engagé en faveur du transport combiné, et à investir fortement dans les ports français, comme M. le Premier ministre l'a annoncé lors du CIMer, au Havre, le 21 janvier dernier. Il faut aller plus loin en dotant les ports français de nouveaux outils juridiques et fiscaux. Les zones franches portuaires peuvent être un levier pour maintenir nos ports à flot. Elles permettent de libérer les marchandises des formalités douanières lourdes et d'inciter fiscalement le transport maritime.

quand pourrons-nous expérimenter les ports francs en France, notamment sur la côte normande ?

Pour rappel, les dépenses de ces touristes britanniques séjournant en France s'élèvent à 1,5 milliard d'euros par an. Par le biais de la TVA, l'État en récupère une part non négligeable, estimée à 250 millions d'euros. Avec la crise sanitaire, les confinements successifs et le Brexit, les entreprises de transport assurant les liaisons entre la France et la Grande-Bretagne sont fortement touchées. Cette situation a des conséquences négatives majeures et entraîne une désorganisation des échanges maritimes sans précédent. L'impact financier sera très lourd, et les pertes de chiffre d'affaires significatives. Entre 2019 et 2020, Brittany Ferries a perdu 70 % de ses passagers-

Désormais, nous devons anticiper sur la sortie de crise et fixer un cap clair pour aider ces entreprises à se relever dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Madame la ministre, avez-vous l'intention de mettre en place un plan de relance spécifique, tant attendu par les entreprises de transport et de service maritime trans-Manche ? Mieux vaut répéter que contredire. C'est pourquoi, pour faire face à une concurrence internationale impitoyable, à la veille d'une saison touristique estivale que l'on espère réussie, ce soutien devrait, me semble-t-il, se traduire par la prise en charge par l'État des charges sociales des personnels des entreprises assurant les liaisons trans-Manche, ainsi que par des campagnes de promotion de nos territoires auprès du public britannique. La

Cette activité, qui assure habituellement le transport de plusieurs millions de passagers chaque année et emploie directement des milliers de salariés, présente un intérêt stratégique et économique majeur pour le pays et pour le département de la Manche. Ses débouchés créent des milliers d'emplois et sont essentiels pour le développement économique du Grand Ouest. Déjà mis à mal par la très longue incertitude due aux négociations du Brexit, le transport trans-Manche a été fortement affecté par la crise sanitaire, qui a fait fuir les voyageurs. À cela s'ajoutent les distorsions de concurrence, qui perdurent, avec les pavillons étrangers. En effet, En effet, les concurrents britanniques sont dispensés de cotisations sociales salariales, et les opérateurs danois se voient rembourser les cotisations sociales patronales et salariales. Si de telles mesures sont licites au regard du droit de l'Union européenne, l'État français n'y a pas recours. Nos opérateurs, à cause de ces coûts salariaux excessifs, sont en position de fragilité, laquelle n'est pas liée au niveau des rémunérations nettes mais véritablement au poids des cotisations sociales dans notre pays. Depuis la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, la route classique pour rejoindre l'Irlande par le tunnel sous la Manche, puis la traversée de l'Angleterre, étant moins rentables, de nombreux transporteurs se tournent vers le port de Cherbourg où des liaisons directes sont assurées vers l'Irlande, ce qui accroît l'activité du port. Cependant, il ne faudrait pas que l'augmentation du fret à Cherbourg soit un feu de paille. Une reprise du trafic à travers l'Angleterre pourrait avoir lieu lorsque les entreprises se seront habituées aux nouvelles procédures. Il nous faut dès maintenant renforcer notre compétitivité et mettre en place une véritable stratégie proactive.

pour la réplique. Le Brexit a mis l'économie de nos territoires de la Manche, de la Normandie et du Grand Ouest en grande difficulté économique, aussi bien le secteur de la pêche, que vous connaissez, que le transport trans-Manche. Nous espérons que l'État français et les collectivités- je suis d'accord avec vous sur ce point -sauront accompagner ces territoires littoraux afin qu'ils ne subissent pas davantage une situation indépendante de leur volonté.

qui devraient donner un autre visage à cette France maritime et terrestre.